j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2022 ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement et la parole est à madame daphné Ract-Madoux pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci madame la présidente, celle-ci concerne scrutin numéro 51 au Plfss pour 2023 notre collègue Jean-Marie Janssens souhaitaient voter. Pour je vous remercie, merci acte donné de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés l'ordre du jour appelle l'examen de 3 projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales pour ces 3 projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifiée,

alors qui est pour, qui est contre qui s'abstient le projet de loi est adopté, je mise aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour, qui est contre qui s'abstient le projet de loi est adopté, je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la déclaration relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour, qui est contre qui s'abstient le projet de loi est adopté définitivement. l'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution en application de l'article 34 ans, de la Constitution, portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France et l'amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre, présenté par Monsieur Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues dans la discussion générale, la parole est au président Guillaume Gontard, auteur de la proposition de résolution et pour dix minutes chers collègues. Avant que vous ne preniez la parole madame la Ministre, Michel, mes chers collègues, les chronomètres sont en panne, c'est pas pour ça que vous allez pouvoir parler tout le temps, monsieur le Président, alors les services sont mobilisés pour les remettre en état de marche en attendant, nous utiliserons des chronomètres Manuel et je vous avertirai en cas de dépassement de votre temps de parole Monsieur le Président, maintenant c'est à vous. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de satisfaction que je défends aujourd'hui devant le Sénat, cette proposition de résolution initiée par le groupe écologiste et cosigné par plus d'une cinquantaine de collègues de tous les groupes de la Haute assemblée et que je remercie une nouvelle fois vivement cette résolution vise à encourager le développement de la filière chambre et à clarifier la réglementation des produits issus du Champ, cela aura été l'un des six le rouge de mon mandat à Paris comme comme en Isère depuis ma participation à la mission sur les bords, l'herboristerie de notre estimé collègue Joël Labbé, en 2018 jusqu'à l'accueil dans nos murs de la 2ème rencontre de l'interprofession du chanvre au mois de mai dernier, entre temps, l'Assemblée nationale s'est saisi du sujet pour produire une mission d'information hors norme, la réglementation environnementale vingt vingt a été adopté, faisant la part belle aux matériaux biosourcés la réglementation un camp près incompréhensible sur le CBD a défrayé la chronique judiciaire, je suis donc heureux de la place que prend la filière chambre dans le débat public et des progrès accomplis, même si beaucoup reste à faire et c'est tout l'objet de cette résolution, qui invite le gouvernement à accompagner cette filière indispensable pour la transition écologique et à clarifier une bonne fois pour toute la réglementation sur le CBD, mes chers collègues me pardonneront si je répète ce matin, certains éléments de mon propos, du 3 février dernier, c'est d'ailleurs ce débat en séance demandée par notre groupe août était apparu une large majorité le majorité de vue sur cette problématique qui a initié la présente proposition de résolution, mais nous avons choisi en en lien avec les acteurs de la filière, de ne pas évoquer uniquement l'imbroglio juridique autour du CBD, mais d'évoquer toute la filière qui même si elle se porte bien, mérite toute l'attention du gouvernement, je le disais en février depuis l'Antiquité, le chambre a pourtant continuellement habillés, nourris, soignés, les hommes et recueilli leurs écrits, aujourd'hui il fait encore tout cela mais pas que il nous loge et peut représenter un substitut au plastique les débouchés industriels sont considérables, mais largement sous-exploité, la France est le 3ème producteur mondial de chant, le 1er européen avec seulement 22000 hectares les surfaces cultivées ont triplé depuis 10 ans et devrait doubler ces 5 prochaines années, rappelons que la culture du chanvre ne suscite pas de produits phyto-phytosanitaires ni d'irrigation qu'elle restructure et dépolluer les sols et s'inscrit donc opportunément dans les rotations de culture. Mieux, elle capte plus de carbone à l'hectare que la forêt 15 tonnes par an, le chambre est informé d'une formidable opportunité pour nos agriculteurs en bio, comment conventionnelle a à condition de multiplier ces débouchés et ça tombe bien, ils sont nombreux, et toute la plante et valorisables, les fleurs et les feuilles Servent à produire le CBD ou à extraire des arômes pour la parfumerie ces graines très riche en protéines, nourrissent l'humain comme le bétail et les animaux avec Loisel, riz, la pêche, la paille permet avec ses fibres de faire de la fibre textile de l'isolant thermique du Bioplastics et des papiers spéciaux et avec son corps solide, la chaîne vote de faire du béton végétale et de la litière s'agissant du CBD je laisserai mon collègue, Thomas Dossus, préciser les choses, nous demandons au gouvernement de ne pas attendre le jugement du Conseil d'État pour autoriser la vente au détail des fleurs, des feuilles du catalogue autorisée que nous proposons d'élargir à toutes les variétés contenant moins de 1 % de THC on est actuellement dans la réglementation à 0,3 pour 100 des milliers d'acteurs économiques attendent la fin de cette mauvaise comédie judiciaire ce flou juridique, mais c'est toi est souhaitable pour personne, nous avons besoin de règles claires facilement contrôlable et d'un encadrement adapté à la fois dans la production du Champ sa transformation et son utilisation pour favoriser les contrôles, nous demandons la cartographie de toutes les cultures de chant, même celles ne faisant pas l'objet d'une déclaration dans le cadre de la PAC les agriculteurs et la filière le demande, nous proposons également, comme en Suisse, d'équiper nos forces de l'Ordre de tests portatif, père de me permettant de mesurer très rapidement le taux de THC de la fleur et de déterminer donc sa légalité s'agissant du volet alimentaire l'arrêté de décembre 2021 ne règle pas toutes les questions posées par la consommation de CBD vous invitons donc le gouvernement à définir les doses journalières recommandées de CBD à exclure de la réglementation novel Food, les produits qui ne sont pas enrichis en CDD et à définir clairement clairement les produits issus du chanvre qui relève d'une consommation de bien-être et pas du régime de la pharmacopée, s'agissant de la filière textile qui a, rappelons-le, un impact carbone 5 à 8 fois supérieur inférieur pardon et consomme à minima, 2 fois moins d'eau que le coton, parfois beaucoup plus, c'est c'est variable bien sûr en fonction des des climats, nous sommes en train de passer un cap avec une réglementation européenne plus exigeante sur l'origine d'Aix textile et avec l'engagement de grands industriels du vêtement pour utiliser justement la fibre de chambre mais les lignes de production et les outils industriels qui travaille la fibre de coton ne sont pas toujours adaptés à la affiche de chambre et demande des réglages important, il faut donc procéder à de lourds investissements pour lequel nous demandons à la puissance publique d'accompagner les efforts engagés par les industriels nous pensons notamment crédit France 2030, qui n'ont pas été intégralement consommé et qui, au delà des technologies de rupture chère au président de la République doivent aussi financer le retour à des savoir-faire ancestraux quand ils sont aussi bien adaptée aux défis écologiques en s'appuyant sur la nouvelle réglementation européenne, sorte de Nutri score des textiles, nous invitons également le gouvernement à mettre en place un Label textiles bio-sourcés et ensuite à l'utiliser dans les critères environnementaux de la commande publique, s'agissant des bio-plastiques qui équipent principalement les tableaux de bord des voitures, je rappelle qu'il est un peu un peu plus un peu moins, par contre, pardon, de 30 % plus léger, recyclable cette fois et que sur le parc de 13 millions de véhicules équipés, ils représentent une économie de 100000 tonnes équivalent CO2, le gouvernement devrait aussi le considérer davantage dans son soutien aux filières industrielles vertueuse, les films de change peuvent aisément remplacer les fibres de verre dans nos nombreux composite et faciliter le recyclage des études sont d'ailleurs en cours, notamment pour la réalisation des pales d'éoliennes s'agissant du bâtiment, il nous faut concentrer nos efforts tant le chanvre répond aux exigences de la transition et rénovation énergétique et limite nos dépendance aux hydrocarbures au mois de septembre j'ai visité une des premières entreprises proposant des modules préfabriqués en béton, le Champ de la chaîne : vote de la chaux Dubois et vous avez un mur qui stockent 35 5 kilos de carbone au mètre carré Quentin béton classique et mais lui 126 kilos de CO2 au mètre carré, vous avez une hygrométrie inégalée qui nécessite extrêmement peu de chauffage et de climatisation 70 % d'économie suivant le CEREMA d'économie d'énergie, évidemment, vous avez un mur biodégradables ou recyclables qui n'est pas un détail : quand le bâtiment est responsable de 3 cinquièmes des déchets du pays pourtant il reste encore des blocages réglementaires, notamment avec les règles professionnelles, le béton de chanvre et plus qu'adaptées aux exigences de la réglementation environnementale vingt vingt il faut massifier son développement et pour se faire former les architectes tous les métiers de la construction, ainsi que les accompagnateurs rénovent ou les conseillers de l'Lana à l'utilisation des matériaux biosourcés et grâce à la laine de chanvre, le secteur de la rénovation comme du neuf d'ailleurs, et de la rénovation thermique n'est pas en reste actuellement 90 % des matériaux du bâtiment sont issus de la filière pétrolière ou minière et leur transformation et considérablement énergivores, selon une étude de l'Ademe, le polystyrène utilisé en une isolation émet de 8 tonnes de CO2 par tonne produite alors que la laine de champs permet-elle de stocker à l'inverse du carbone est également recyclables et biodégradables ainsi en cohérence avec la réglementation environnementale vingt vingt nous invitons le gouvernement a fixé des critères ou des bonus pour les aides à la rénovation thermique MaPrimeRénov'éco-PTZ en lien avec la performance environnementale des matériaux utilisés, au passage, cela vaut pour le chanvre et tous les matériaux beau sur succès et je vous annonce en exclu visite et lui éviter un amendement écologiste au PLF en ce sens, tout juste déposé sur le prêt à taux 0, une fois que j'ai dit tout cela, vous l'aurez compris il faut massifier la culture et l'utilisation du et cela passe peut passer notamment pas par une grande campagne de communication publique à destination des collectivités, des professionnels et du grand public, promises notamment en 2018 par le plan d'action une stratégie bioéconomie pour la France, mais jamais pour l'instant mise en oeuvre, néanmoins, nous sommes inquiets sur les capacités de production agricole pour 2023 la guerre en Ukraine a tellement fait exploser les prix des grandes cultures, notamment des céréales que nos agriculteurs n'ont pas d'incitation financière à planter du chanvre cette année en 2023 à l'hectare, le chanvre rapportera 20 100 de moins que le maïs, le blé ou colza aussi la filière nous formule une demande supplémentaire qui n'était pas saillante au moment de la rédaction de cette PPR mais qui nous semble, au combien légitime la reconnaissance sur le marché carbone réglementés du carbone stocké par l'ensemble de la filière, j'ai, je le crois suffisamment détaillé le bilan carbone phénoménal de la culture et de l'usage du chance pour vous convaincre du bien-fondé d'une telle demande pour cela, la filière a demandé un accompagnement de la part des corps d'inspection de l'État afin de créer un mécanisme de reconnaissance du stockage du carbone au bénéfice des producteurs car les spécificités de la filière chambre profondeur racinaire poursuite du stockage de carbone dans les débouchés sont mal prises en compte par le modèle créé par le Label bas-carbone la stratégie nationale bas-carbone pourraient également être renforcée par une prime au stockage de carbone dans la rénovation thermique des bâtiments pour notamment inciter l'utilisation d'isolation biosourcés il conviendrait enfin de favoriser les matériaux biosourcés grâce à la réduction de la TVA et on compte sur le gouvernement pour obtenir cette satisfaction à Bruxelles, dans le cas de la refonte de la directive TVA voilà, mes chers collègues, une présentation succincte et que notre collègue dessus complétera de l'armée américaine, si pour d'approbation du Sénat afin d'envoyer ça va mais respecte au gouvernement et mettre davantage en lumière et filières pleine de promesses dans bien des territoires notre vote est attendu par des centaines d'acteurs économiques

je on passera pas la matinée et il y a des personnes qui ont des d'autres choses à faire derrière, donc je vous demanderai de vous respectez les uns et les autres, merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes chers collègues.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui permet donc de mettre en lumière une filière parfois méconnus du grand public, à ce titre, je salue cette initiative qui permet ainsi d'évoquer un sujet d'avenir sur le plan économique pour nos territoires, la filière du Champ, l'opinion publique, ce patient généralement pour les découvertes qui marque une rupture avec leur temps, à l'inverse, l'exemple du chanvre est symptomatique d'un réel engouement pour une redécouverte. En effet, si le sujet ne prend de l'ampleur que depuis quelques années, son utilisation par l'être humain est multiséculaire, alors évidemment, et puis il y pas de méprise l'évocation du chance fait souvent penser au cannabis est souvent associé à la triste réalité du trafic de drogue et de ses conséquences dramatiques, notamment chez les jeunes, je pense que la première des priorités sur ce sujet, donc un travail pédagogique, il faut bien distinguer le drame que constitue le cannabis utilisé comme drogue et la filière chanvre qui apparaît comme une formidable opportunité dans de nombreux domaines économiques le chanvre est une plante qui permet de stocker le carbone c'est une plante qui a un bilan carbone formidables qui nécessite peu d'énergie, peu d'intrants et peu d'eau pour sa production, elle peut s'utiliser dans le secteur du bâtiment de la commission de la cosmétique de l'alimentaire ou encore dans le textile. Pour ce qui est du secteur du bâtiment le crépi chaud chanvre en intérieur, sur du bâti ancien ou récent permet d'éviter l'usage de la climatisation, le show chambre absorbe l'humidité pendant les périodes froides et le restitue en période chaude, alors que la sobriété énergétique s'impose comme une priorité nationale, le chanvre, constitue une véritable alternative à nos modes de fonctionnement traditionnels, la nouvelle réglementation environnementale les bâtiments neufs, la R 2020, va dans le bon sens puisqu'elle met en avant les matériaux biosourcés néanmoins certains verrous réglementaires pourraient être levées ou améliorer, on pourrait ainsi imaginer la prise en compte d'autres critères que le coefficient thermique comme les polluants ou encore le confort de vie, il pourrait également être pertinent de mieux accompagner financièrement la production, l'usage des matériaux biosourcés. Compte tenu de l'envolée des prix des matières premières, le apparaît également comme un substitut formidables pour remplacer la laine de verre, la laine de roche ou encore bien sûr le polystyrène, enfin, il existe un véritable défi autour de la formation des professionnels du bâtiment afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'utilisation de la fibre de chanvre dans les auditions des combles et des parois des bâtiments mais également dans l'usage de la chaîne votre dans les crépi isolant, il est fondamental d'informer les décideurs publics de ces formidables atouts autre exemple dans le département de la Charente-Maritime qui m'est cher, le projet de territoire pour la gestion de l'eau de la rivière de la boutonnent travaille sur plusieurs axes, à savoir les aspects qualitatifs et quantitatifs de l'eau ainsi que sur celui de la protection des milieux de plus, il y a une véritable volonté locale de trouver une culture de n'assistant pas de pesticides ne n'Systems nécessitant un minimum d'engrais, tout en dégageant revenu correct pour les producteurs, au delà d'apparaître comme une solution intéressante la filière chambre demeure la seule solution pouvant répondre à l'ensemble de ces critères. Il y a également, bien sûr, une filière alimentaire du Champ grâce à l'utilisation à la transformation des graines de chanvre en huiles tourteaux farine ou encore chocolat à une époque où le circuit court est plébiscité par nos compatriotes le chance permet de répondre à ces nouveaux modes de consommation, la filière textile est encore trop peu développée par rapport à son potentiel, je rappellerai à ce titre que le jeans denim était historiquement produit à partir de chambre avant d'être en coton, au moment où la rémunération des agriculteurs soulève souvent un émoi légitime dans l'opinion publique cette filière apparaît aussi comme source de rémunération très correct pour les producteurs, c'est donc un levier économique qui vient compléter cette formidable palette de plus caractéristique du chant. Enfin, alors que nous venons d'examiner en première lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, je tiens à saluer la prolongation de l'expérimentation du cannabis thérapeutique, nous sommes encore au au stade embryonnaire, côté prescription sans c'est un vrai statut de médicament mais dont l'intérêt médical est particulièrement encourageant pour toutes ces raisons, le bâtiment une liquidation dans le bâtiment, dans l'alimentation dans le textile en médecine pour toutes ces raisons et en souvenir des cordages de chant fabriqué à la Corderie royale de Rochefort sur Mer à titre personnel, je voterai cette proposition de résolution, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Vanina Paoli-Gagin. Pour le groupe, les indépendants pour cinq minutes chers collègues.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution est une excellente opportunité de parler d'une filière chambre à la fois complexe et prometteuse complexe car elle regroupe de nombreux acteurs de toute taille et concernent finalement des industries très diverses, ce qui fait la force, mais aussi la faiblesse prometteuse aussi, et ce à plusieurs égards la France est le 1er pays, ça a été dit, producteur de chanvre en Europe, mon département de l'Aube, très à la pointe sur cette filière produit près de 50 % de la production française, un tiers de la production européenne nous développons cette culture depuis des décennies sur ce territoire à forte tradition industrielle, la maison de la Turquie à Nogent sur Seine bâtissent toutes Flaubert, Sienne a été rénové avec des béton chanvre, l'industrie du bâtiment place de grands espoirs dans les matériaux de construction à base de chanvre, industrie textile très polluantes se tournent aussi de plus en plus faire ce matériau à l'heure où la mode éthique, c'est entrer dans les consciences, la nécessité de changer la donne, plus largement, l'utilisation du chanvre dans certaines industries participe activement de notre transition vers la neutralité carbone cette culture, cela a été dit, n'a pas besoin de beaucoup d'intrants, elle est très peu consommatrices d'eau, ce qui limite les besoins d'irrigation, c'est un atout agro-écologique majeur dans le contexte du réchauffement climatique que nous connaissons le chanvre à la capacité de stocker beaucoup de CO2, cela a été dit également par mes collègues dans un laps de temps très court, absorbe sur une année environ 15 tonnes de CO2, c'est-à-dire que c'est exactement le même montant que ce absorbe un hectare de forêt le chanvre et donc une culture aux multiples externalités positives, notamment pour les soldes dans le cadre des rôles des rotations culturales, des atouts cruciaux pour notre agriculture, mais pour que cette chance se transforme en marché, encore faut-il des débouchés stables pour la filière, bien sûr, les investissements sont indispensables, être au fait des réalités du secteur nous permettra de gagner en compréhension et donc d'agir en conséquence, d'après la proposition de résolution dans 5 ans, cette filière pour créer autour de 20000 emplois et représenter un chiffre d'affaires annuel qui avoisinerait les 2,5 milliards d'euros, la France doit transformer l'essai. Je pense que la poursuite du développement de cette filière participera à la réindustrialisation de notre pays, à laquelle je suis très attaché, nous devons continuer à nous battre pour faire émerger des champions industriels et j'en profite pour saluer les annonces récentes du ministre délégué chargé de l'industrie sur les stratégies de relocalisation industrielle et le produire en France dans nos territoires, je pense que la filière chambre peut servir si ces impératifs, nous avons de l'avance et pourtant nous devons aider à structurer cette filière,

c'est là qu'intervient l'importance des matériaux biosourcés et de leur développement à ce titre-les points 30 31 et 32 de la proposition de résolution sont très intéressants, les matériaux biosourcés ont toute leur place dans nos démarches de rénovation et de lutte contre les passoires thermiques, nous devons faire en sorte de mieux faire connaître ses produits à la fois des professionnels mais aussi de nos concitoyens, j'aborderai un dernier point : celui du CBD dès janvier, j'ai posé une question au gouvernement sur l'avenir de la filière après le fameux arrêté du 31 décembre 2021 oui une régulation est nécessaire et la filière n'y est pas opposé la proposition de résolution met en lumière les chiffres des millions de consommateurs ainsi que des milliers de points de vente, les acteurs auront besoin de stabilité, je le répète, la position de la Cour de justice de l'Union européenne, celle de l'OMS également s'inscrivent dans une même optique le CBD n'est pas un stupéfiant avec ses taux de THC inférieure à 0 3 % là encore, Madame la Ministre : Ne laissons pas nos voisins européens, affaire Tapie sur le marché français s'il vous plaît, avançons ensemble dans un cadre qui respecte à la fois la santé publique et qui permettront à nos entrepreneurs d'innover en revanche certains points dans cette proposition de résolution me semble plus problématique, je n'ai malheureusement pas le temps de les détailler, mais je ne suis pas sûr de la pertinence de la multiplicité des labels qui sont proposés, le point 26 concernant l'élargissement du catalogue cultivars variétés qui contiennent moins de 1 % de THC m'interpelle également toutefois et pour toutes les raisons énoncées ci-avant notre groupe les indépendants dans sa majorité votera en faveur de ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Thomas Dossus. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires et pour cinq minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en introduction, le président Gontard vous a présenté le potentiel de la filière française du change d'un point de vue industriel je voudrais de mon côté, me focaliser sur un produit particulier de cette filière, le CBD mais en préambule, tant la confusion peut parfois régner un effort de définition s'impose lors que l'on parle de chambre de CBD ou de THC, on parle de la production de 2 espèces de plantes très proches biologiquement si le sang une un produit issu du traitement de la fibre de ces plantes le CBD ou cannabidiol et le THC, le tétrahydrocannabinol sont des des molécules provenant de fleurs, lorsque l'on parle de cannabis récréatif, on parle du THC alors rappelons-le pour éviter tout amalgame le CBD n'a strictement rien à voir, nous parlons bien de de molécules différentes, avec des effets différents si le THC est considéré à juste titre comme un psychotrope, avec tous les risques d'addiction, d'un point de vue médical le CBD n'engendre pas d'addiction et les effets psychotropes sont inexistants, à ce titre, il n'est pas recherché lors des tests de dépistage des stupéfiants par les forces de l'ordre, lorsque l'on parle de CBD en tant que produit commercialisé, on parle d'extraits de fleurs de chanvre que certains trouvent apaisant antistress présentant un taux de THC inférieur à 0 2 % c'est-à-dire très très largement en dessous du seuil à partir duquel se manifeste les effets psychoactifs pourtant une certaine confusion existe parfois dans les esprits et lorsque l'on regarde l'évolution de la législation autour du CBD, on constate que cette confusion règne jusqu'au sommet de l'État, et ce dès l'apparition de la filière en France, au grand dam de notre filière agricole les premières boutiques de vente de CBD apparaissent dans notre pays en 2018 et certaines seront fermées régulièrement par la police en raison d'une mauvaise interprétation d'un arrêté de 1990 daté et inadapté à ce nouveau marché. Pour y remédier, en juin 2018, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives à la brillante idée de distinguer le CBD synthétique du CBD récolté naturellement, sans même mentionner le côté scientifiquement inepte de ces distinctions, celle-ci mais alors la France en situation de non-respect du droit communautaire européen non respect, confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne en novembre 2020 en raison d'une entrave au principe d'égalité devant la loi et de la et de libre échange au sein de l'Union, le gouvernement a pour y remédier, une nouvelle idée encore plus brillante qui prend, arrêté en décembre 2021 autorisé le CBD en tant que molécules mais interdire la commercialisation de la fleur de chambre, ainsi que son utilisation en infusion ce nouveau trait de génie administratif bien français ne mettra pas longtemps à recevoir son jugement mérité une suspension par le Conseil d'État, en janvier 2022 le jugement au fond est encore attendu. Ces 2 décisions du gouvernement, témoin, bien qu'il y a là un malaise, une confusion, une instrumentalisation de la filière CBD dans des buts moraux et une forme de déni de la science, nous le disons et nous le répétons-le CBD n'est pas une drogue, même s'il contient des traces infimes de THC, il faut cesser d'urgence cette confusion entretenue à dessein, car des emplois une filière agricole et industriel ainsi que commercial sont en jeu, 1800 boutiques spécialisées, plus de 30000 emplois si on prend en compte la production, la distribution, la commercialisation pour satisfaire la demande de 7 millions de consommateurs tous ces commerçants vivent dans une grande insécurité à cause de revirements réglementaire et craignent pour leur avenir, si au contraire on en finissait avec cette confusion permanente et que l'on soutenait réellement la filière on pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires le CBD n'est ni une drogue ni un produit addictif, il est utilisé, il est utilisé dans toutes les tranches de la société et à tous les âges, les Françaises et les Français aiment ça, madame la Ministre, finissons en avec la confusion permanente et revenons à la science qui fait bien la distinction entre les 2 molécules ETH et le CBD permettons l'essor de toute une filière composée d'employes locaux et de commerces de proximité, le pouvoir réglementaire est entre vos mains, utiliser utiliser le à bon escient Merci monsieur dossier, la parole est à madame Nicole Duranton. Pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour six minutes chers collègues. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, lorsqu'on additionne toutes les vertus du chanvre, on ne peut être que conquis aucune autre plante ne semble cumuler autant d'avantages ne coche autant de cases environnemental et économique, nous sommes tous d'accord, ça a déjà été dit par mes collègues le chanvre c'est d'abord une plante qui consomment peu d'eau au sortir d'une année marquée par la sécheresse et alors que la question de la préservation de la ressource en eau et de plus en plus problématique, c'est un atout considérable notre climat est particulièrement propice à son développement, un développement qui est rapide, puisqu'entre la graine et la récolte, il ne s'écoule que 4 mois avec un rendement maximal, une plante qui n'a pas besoin d'herbicides, de fongicides et d'insecticides, là encore, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la ressource en eau, puisque cette plante n'a pas besoin pour se développer, de polluer les nappes phréatiques, avec des traitements ou des intrants chimiques autre atout cette plante est aussi tout indiquée dans leur rotation des cultures régénèrent la terre et permet sur la culture suivante un gain de rendement de 5 à 10 % pour les céréales, enfin le chambre est aussi un excellent pièges à carbone puisqu'on considère qu'un hectare de chanvre absorbe au moins autant de CO2 qu'un hectare de forêt le chanvre a aussi l'Avantage d'intéresser de multiples secteurs, ce qui lui garantit de nombreux débouchés et là encore, mes collègues l'ont déjà dit dans l'alimentaire, les graines de chanvre et l'huile de graines sont des compléments alimentaires reconnu pour l'humain, comme pour l'animal dans l'industrie cosmétique de nombreux produits utilisent de l'huile de graines de chanvre, dont les vertus sont connus dans le bâtiment, la laine de chanvre et l'un des isolateurs naturels les plus efficaces, le béton de chanvre est également de plus en plus reconnue pour ses qualités naturelles dans l'industrie automobile le la et le Champ ont beaucoup de propriétés commune, on les retrouve d'ailleurs dans les matériaux composites dans l'industrie textile les tiges de chambre possède une forte résistance pour en faire des vêtements et des cordages, dans mon département de l'Eure, la coopérative de l'un du Neubourg vient d'inaugurer une toute nouvelle usine de teillage, la French filature, c'est une petite révolution dans le milieu textile en effet la Normandie Terre de Lin détient la moitié des surfaces de culture en Europe mais elle n'avait plus aucune filature le, l'un étant systématiquement expédiés vers l'Asie avec cette filature, on peut désormais produire du lin, 100 pour 100 tracé Made in France pour l'habillement cet investissement de 5 millions d'euros va permettent de produire plus de 250000 tonnes de fil de lin par an et pourrait parfaitement demain servir pour filer le chanvre en Normandie, il y a un véritable enjeu avec 10500 agriculteurs qui ont plus de 60 ans et qui se prépare à partir en retraite d'ici 2028, autrement dit un agriculteur sur 3 va arrêter et doit être remplacé la culture de chanvre pourrait constituer un marché extrêmement prometteur et ouvrir de nouveaux horizons à nos agriculteurs et même motiver les plus jeunes à s'installer ou reprendre les exploitations familiales en fait cette plante n'a qu'un inconvénient, mais pas des moindres, il faut maîtriser illimité, son taux de THC cette substance psychotrope qui permet de la différencier de la marijuana, en dépit des propriétés formidables de cette plante de ses nombreuses applications et de toutes ces ces, ces perspectives prometteuses, il nous faut donc faire preuve de prudence sur les produits de consommation à base de Cana bidule en effet le CBD n'est pas classé comme un stupéfiant, mais il s'agit tout de même d'une substance à effet psycho actifs dont les risques pour la santé des consommateurs n'ont pas encore été complètement évalué malgré la pression de tout un secteur et le fait que ce sont les cultivateurs de change de pays étrangers qui profitent aujourd'hui de notre marché intérieur, nous devons approfondir nos connaissances scientifiques sur le CBD avant de délimiter un cadre législatif le CBD est aujourd'hui autorisé à la commercialisation en France mais des progrès doivent être faits pour mieux contrôler les produits qui sont aujourd'hui mis sur le marché, la filière qui voit dans ce débouché bien être une opportunité de développement poussent notamment pour établir des normes pour procéder à des contrôles de teneur mais aussi encadrer les méthodes d'extraction et d'analyse et fixer des seuils réglementaires transitoires ce sujet technique mais il est fondamental et ne supporte pas l'approximation, en effet, lors de l'extraction du CBD de la plante, il y a un risque de concentrer aussi l'extrait en THC si l'extraction et mal maîtrisée, or celui-ci a un seuil de toxicité aiguë très faible, une réflexion interministérielle est en cours visant à délimiter le cadre d'une politique de contrôle pour écarter du marché les produits les plus problématiques la PPR propose d'ailleurs des orientations intéressantes sur ce point qui mérite d'être approfondie, le ministère de la Santé, s'interroge sur la toxicité du CBD et le ministère de l'Intérieur sur son caractère addictif, le F. S. à l'Autorité européenne de sécurité des aliments procède actuellement à des évaluations plus précises du CBD et nous gagnerons sans nul doute à définir nos politiques publiques sur la base de ces données scientifiques affiner, même si les résultats de ces études ne seront pas connus avant plusieurs mois, par ailleurs, il faut être attentif à ce que le développement de la filière CBD par sa rentabilité n'assèche pas mécaniquement les autres débouchés qui sont porteurs de souveraineté alimentaire ou énergétique pour toutes ces raisons, notre groupe, le RDPI s'abstiendra je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gilbert Luc devina pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes. Merci. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si la culture du chanvre accompagné l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps, cette plante a bien failli disparaître au XXe siècle avec l'arrivée de la pétrochimie, la France est resté le seul pays à maintenir sa production, c'est pourquoi elle est leader sur le marché européen aujourd'hui. La nécessité de produire 100, sûre, durable et accessible. Tous remet cette plante au goût du jour, elle répond parfaitement aux attentes sociétales et environnementales sans produits phyto-pharmaceutiques sans irrigation sans OGM, le chanvre. étant réservoir à à biodiversité et absorbe autant de CO2 que la forêt, la filière est 100 % française de la sélection variétale à la transformation de plus, les produits qui en. Sont issus sont compostable et recyclable en fin de vie, toutefois cette culture nécessite beaucoup de travail, avec souvent de 4 à 7 passages et un matériel spécifique, très coûteux, c'est donc la récolte qui est un frein au développement du chambre auprès des agriculteurs, le chanvre est éteint probablement la plante la plus polyvalente connus de l'humanité, elle n'est malheureusement connue du grand public que par sa fleur dans le secteur du bâtiment. Le recours aux chambres est en expansion depuis plusieurs années du fait de ses qualités en terme de régulation thermique de résistance au feu ou de légèreté l'inter-profession se fixe aujourd'hui comme objectif majeur : la construction du village olympique de Paris 2024 avec le chambre : le recours à la paille et. Fibre de lin et de chante sera notamment accrue accrue et pourrait donc présenter un débouché important une vitrine médiatique forte pour la filière avec la délégation. Si aux entreprises nous avons visité dans le département du Rhône, en mars dernier l'entreprise si ma. Vicat à Feyzin, située dans la vallée du Rhône, sur la métropole de Lyon la solution débloque de chambres emboîtement de Vicat a été primé par l'institut français pour la performance du bâtiment cette solution brevetée met en oeuvre des granulats de chèvre chez vos notes et un Vian à base de ciment qui lui confère des porteurs moment s'exceptionnel. Un débouché important pour ce secteur qui se renouvelle totalement la culture du chanvre. Peut présenter l'un des piliers de notre réindustrialisation écologiquement responsable, qu'il s'agisse de filières de construction locale, s'appuyant sur la culture durable du chambre et du qu'il s'agisse des industries textiles locales beaucoup plus économes en eau et en intrants que l'industrie du coton, qu'il s'agisse du développement des bio-plastiques plus léger et compostable qu'il s'agisse d'une filière papier réinventer, qu'il s'agisse du développement des protéines végétales pour diversifier notre alimentation, qu'il s'agisse des industries co-mystique pharmaceutiques et du bien-être aussi je. Poursuite de ce texte pour souligner que cette filière à usage industriel n'a pas bénéficié du plan de relance, car ces projets n'étaient pas prêts, or l'accompagnement de l'État est nécessaire pour la massification industriels de cette filière, cette dernière. L'Avantage d'être en phase avec les objectifs de neutralité carbone de la France, tout en étant une industrie au savoir-faire local bien implantés territorialement dans le secteur Tessier textile de chambre est une solution écologique qu'il est urgent de développer pour transformer le modèle de production pour cela les investissements industriels conséquent sont nécessaires, la rémunération des producteurs est également un enjeu majeur pour permettre

et la dynamique de cette filière soit reconnue, il faut également accompagner le développement des matériaux biosourcés dans le cas de la rénovation énergétique des bâtiments formés, informer, inciter le chambre doit donc être au coeur de la relance de notre économique pour accroître nos sous souveraineté renforcer nos territoires et réduire les impacts environnement manteau de nos activités. Qu'attendons. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste. Républicain citoyen et écologiste pour cinq minutes. minutes. Ministre, mes chers collègues, le groupe C CRCE votre en faveur de la PPR qui vise au développement économique de la filière chanvre et à l'amélioration de la réglementation des produits issus de ces plantes, tout devrait assurer un développement majeur de la culture et la transformation du chanvre dans notre pays, les collègues l'ont déjà dit, la planter sa culture parfaitement adaptée au climat français peu d'utilisation d'eau et d'entrants pas de de destruction des sols au contraire stockage efficace du carbone, les usages sont variés, vous l'avez dit tissu nourriture bâtiment substitut naturel au plastique et bien sûr des vertus thérapeutiques alors pourquoi de telles opportunités ne se concrétise-t-elle pas, en tout cas pas assez passe une variété de chanvre le cannabis produit des des fleurs, une fleur aux effets psychotropes est considéré comme un stupéfiant et au motif de combattre de cette plante et son usage les réglementations sont restrictives bien au-delà de ce qui serait nécessaire, instable, freinant le développement de cette filière très utilisées pour la transition écologique,

de surcroît, on sait qu'un autre principe actif, comme le cannabidiol, ou CBD a des propriétés apaisantes et dans certains cas même apaiser douleur que d'autres formes de produits n'arrive pas à affaiblir et peut être évidemment issu d'une variété du cannabis, mais d'une variété le cannabis sativa L mais on ne sait pour quelle raison dans un pays de la rationalité, on a instauré une réglementation qui n'était pas cohérente et intelligente avec nos exigences sur la législation contre les stupéfiants et d'autre part sur une capacité à développer l'usage du Champ dans tous les domaines et même pour la consommation de car car soyons clairs, il ne s'agit pas d'ouvrir ici ni de contourner le débat sur la législation du cannabis, c'est un autre sujet, il ne faut pas entretenir cette confusion, or on a plutôt l'impression que chaque fois qu'on ait vu avec ce ce problème on on est, on a les yeux rivés là-dessus comme une sorte d'angoisse alors que, je le répète, il faut avoir une attitude rationnelle qui ne confond pas tout. Donc on a un mot d'abord sur la réglementation du CBD, nos collègues ont déjà expliqué, on l'a mal soit évoqué ici sur les imbroglios les les enjeux, les incompréhensions, moi je vais vous dire une chose, je pense qu'en l'état actuel des de la situation, il faut s'en tenir à la réglementation européenne, les autres pays sont pas plus insouciants par rapport aux risques de santé par au risque de au risque des stupéfiants et il faut donc prendre cette réglementation l'adapter à notre pays de manière claire et en particulier permettent l'usage directe de la fleur et des tisanes de ces, de ces plans car ils ne sont pas stupéfiante, or j'entends bien, nos collègues qui nous explique l'Europe s'interroge sur la révision de cette législation et bah, écoutez, prenons la telle qu'elle est et on évoluera, quand l'Europe aura évolué, ça avait l'argumentaire va attendent l'Europe pour voir comment ça va évoluer, on l'a entendu sur les Gafam, on attend toujours donc je suggère qu'on agisse dans le cas de la législation actuelle et qu'on évolue, le moment venu, ça suppose d'ailleurs qu'on développe et c'est dans la PPR des organes de contrôle, contrôle des tests, il y a des tests maintenant qui sépare les stupéfiants : cannabis et le CBD la teneur en THC, d'autre part, je crois que l'idée d'avoir une cartographie des plantations de chanvre permet premièrement de contrôler ce qui serait pas légal plus facilement et d'autre part d'assumer comment notre filière évolue et si le rendez-vous de de de son développement, alors il y a dans cette PPL évidemment d'autres sujets, ah oui, je voudrais insister 90 % de la consommation du CBD en France qui se développe énormément vient de produits de l'étranger, donc franchement c'est c'est aberrant, hein, et c'est d'autant plus aberrant qu'on passe notre temps à dire qu'il faut regagner notre souveraineté si chers collègues et chers collègues, pour les autres usages du chant, je crois que le consensus est assez large et on aura l'occasion à l'examen des articles de parfois nuancés mercredi. Merci beaucoup, la parole est à madame daphné Ract-Madoux pour le groupe. Union centriste et pour quatre minutes chers collègues. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les multiples qualités du chanvre. Semble faire l'unanimité ce matin et je vais redire peu ou prou ce que vous avez précédemment entendu de mes collègues. Des tout premiers livres imprimés au XVe siècle aux voiles de bateaux qui ont permis de découvrir l'Amérique, le chanvre a eu au fil des siècles le vent en poupe. La culture du chanvre a ainsi discrètement mais sûrement accompagner notre histoire fleur fibre granulés ou chaîne votre la plante sous toutes ses formes est utilisé dans des secteurs aussi nombreux qu'éclectique, l'agriculture, la pharmacie, le BTP, l'alimentation, les cosmétiques, le textile et même Loisel. De 2900 avant notre ère, à la fin des années 30 la culture millénaire du chanvre est alors un impondérable des sociétés humaines le est même qualifié de produits de première nécessité, au même titre que le pain jusqu'au XIXe siècle. Pourtant, peu avant la moitié du XXe, cet âge d'or se termine à la filière dépérit progressivement souffrant de la concurrence des plastiques et de l'amalgame avec la production du cannabis avant de connaître un nouveau souffle dans les années 90 avec mes collègues du groupe centriste nous souhaitons d'ores et déjà être clair à ce sujet, nous voterons ce texte aujourd'hui afin de promouvoir la filière économique du chanvre et le sujet n'est pas ici le THC et le cannabis substance psychotropes, oui, la culture de chanvre est une filière économique d'avenir pour notre pays sous ses différentes expressions, leader européen en la matière, la France peut voir plus grand, la filière doit être à ce titre-pleinement soutenu dans le cadre du plan France 2030, oui, nous pouvons nous appuyer sur le Champ pour contribuer dès aujourd'hui à bâtir notre transition écologique préservant la qualité de nos sols faiblement vorace en eau et requérant peu ou pas de produits phytosanitaires le présente des qualités écologiques évidentes que nous ne pouvons ignorer oui, la culture de chanvre, peut être un atout pour notre agriculture en proposant une diversification des activités et des revenus complémentaires non le chanvre n'est pas portion congrue dans l'équation économique actuel en 2020, cette culture représentaient près de 1414 producteur et environ 30000 emplois Directs et indirects dans mon département, l'Essonne, la culture du chanvre, c'est l'entreprise Gatti chanvre qui travaillent avec près de 100 agriculteur partenaire pour produire 1000 hectares de chanvre dans la moitié en bio. Cette société réalise la première transformation du chanvre, le défi barrage de la paille, cela permet par la suite de production de papier d'isolant de route ou encore de bio-composites, preuve de la variété des productions de la filière, l'entreprise produit exact également de la chaîne, vote qui alimentent les marchés du pays de la litière mais également du bâtiment pour les enduit béton et blocs de chanvre je tiens donc à saluer le travail d'excellence fait par l'ensemble des acteurs du groupe en Gâtinais et maintenant dans les départements limitrophes. à l'aune des à toute cette filière méconnu, je souhaite féliciter nos collègues du groupe écologiste pour la qualité de leur travail sur cette proposition de résolution, loin des clichés éculés de l'inventaire à la Prévert dépourvue d'intérêt, c'est un texte de qualité qui permettent d'alerter les pouvoirs publics sur les changements nécessaires pour développer sereinement la filière cependant, nous devons rester vigilants et nous assurer que nous posons les bases d'une filière souveraine et et coresponsable en construisant des écosystèmes économiques locaux et des débouchés industriels en France, chers collègues, c'est pour cela qu'avec ma collègue Annick Billon et le groupe de l'Union centriste nous voterons ce texte pour développer dès demain avec exigence et ambition la filière chambre je vous remercie. Merci. L'État Monsieur Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues. Il a fallu attendre une décision de la Cour de justice européenne hein 2020 pour que la France autorise en fait les extraits de chanvre et le CDD en tant que molécules mais il faudra encore compter sur le Conseil d'État pour que la commercialisation de la fleur de chambre soit possible, les auteurs de la proposition de résolution le souligner et je tiens à les remercier ces revirements et sécuriser la filière une filière qui compte déjà 30000 emplois Directs et indirects si les aléas juridiques ne cesse pas, la France prendra un retard considérable dans le développement de la culture du chanvre, alors même que notre pays le premier exploitant d'Europe grâce à des conditions climatiques favorables.

mon groupe soutiennent toutes les politiques de lutte contre les addictions aux stupéfiants, la consommation régulière de cannabis mettent en péril la synthétique et psychique, de nombreux jeunes, il est important de le souligner, toutefois, ne nous trompons pas de débat, la législation du cannabis de autre le rappelle, donc, clairement, ce qui nous intéresse à travers ce texte, c'est l'avenir des produits CBD dépourvue d'actifs psychotrope ou contenant moins de 0 virgule il s'agit d'apprécier le large potentiel, le développement du au regard de ses atouts sur le marché, le textile, la construction, le papier ça oublié ses vertus cosmétiques et pharmaceutiques face à cela, comme nous y invite, à la proposition de résolution l'agriculture française pourrait en profiter d'une d'une filière encore plus dynamique, à condition que le gouvernement prenne une position claire et éclairé, mes collègues ont parfaitement présenter les qualités du et qu'on Manon adapté pour la rotation des cultures et offrant une qualité de drainage son exploitation peut donc s'inscrire dans une démarche durable et bénéficier de la belle, comme cela est proposé par ailleurs le développement du chambre peut être dans certains territoires ruraux, un pilier de la reconquête industrielle le RDSE souhaite toutefois posé quelques conditions : la première c'est que son exploitation ne concurrence pas d'autres cultures, essentielles à l'objectif de souveraineté alimentaire que nous sommes nombreux à des fans sur ces bas sa bonne rotation avec d'autres cultures, apporte une première garantie, la seconde condition c'est que sa production et sa commercialisation à des critères de sécurité et de contrôle, l'interprofession se dit prête à un contrôle renforcé des parcelles de champs et à leur déclaration pour la traçabilité des fleurs, je retiens également les propositions du texte quant à la conduite de tests sur les teneurs CBD était HEC, des produits bruts, les flux de marché doivent également être surveillées, pour cela, le développement de la filière doit s'exercer dans un environnement réglementaire sécurisé sur le plan national, comme je l'ai dit, ainsi que sur le plan européen par une uniformisation du taux de THC, le fameux arrêté Kanavape impose au nom de la libre circulation des marchandises à chaque pays, la reconnaissance des teneurs légalement fixée chez ses partenaires, ce qui crée des normes différentes d'un pays à l'autre, cette situation peut compliquer la tâche des services de contrôle, que ce soit la douane et la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, au titre des services, ce que les producteurs de chanvre pourrait rendre à travers le stockage de carbone ou le développement de matériaux biosourcés je souhaite que la mode de la filière soit soutenu, comme le sont toutes les autres, mes chers collègues, la culture du chameau présente un intérêt certain pour notre économie, disons-le aussi, ces produits dérivés répondent à une demande sociétale autour du bien-être, dans ces conditions, la majorité de notre groupe, approuve la proposition de résolution et vous demande, Madame la Ministre, de ne pas laisser la filière perdant pied au profit d'autres pays, mieux préparés, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Laure Darcos ce pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Merci madame la présidente, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de résolution de nos collègues du groupe écologiste qui souhaite alerter le gouvernement sur les contraintes réglementaires pesant sur la culture du chanvre je vous surprendrai certainement ou disons que je partage une partie de leurs préoccupations et de leurs attentes, en effet, le chambre est une plante disposant d'une formidable potentiel d'avenir mais dont les débouchés sont actuellement limitées, pour des raisons dont la logique m'échappe pour nos agriculteurs, elle représente une possibilité de revenus complémentaires, je parle bien de revenus complémentaires car il serait totalement illusoire d'imaginer qu'elles se substituent aux autres cultures pour notre pays, le chanvre, peut être un des moyens d'atteindre une partie de ses objectifs en matière de transition énergétique grâce à son utilisation massive dans le cas de la construction et de la rénovation des logements toutefois la proposition de résolution de nos collègues, met l'accent sur les principes actifs de cette plante et les usages récréatifs qu'elle permet, c'est sa principale faiblesse, or son utilisation dans de nombreux secteurs de l'économie est possible, en particulier dans le bâtiment comme je viens de le souligner, beaucoup de chemin a été parcouru depuis la première rénovation d'une maison d'habitation avec un enduit constitué de chaud et de chambre en 1986 la filière est aujourd'hui parfaitement structurée avec un unique producteur de semences certifiées qui investit puissamment dans l'innovation variétale afin de créer les nouvelles variétés de haute qualité adaptés au marché, l'association construire en chanvre et quant à elle, un acteur majeur pour les professionnels du bâtiment, elle est à l'origine des règles professionnelles exécution d'ouvrages en béton de chanvre qui constitue le 1er et, à ce jour le seul texte de référence sur l'utilisation du chanvre dans le secteur de la construction, dans le cadre sécurisant et sécurisé, de plus en plus d'agriculteurs optent pour cette voie de diversification agronomiques, respectueuses de l'environnement et prometteuse en terme de retombées économiques, mon département, l'Essonne et d'ailleurs l'un des plus importants producteurs de chanvre industriel avec un millier d'hectares en culture et une centaine d'exploitation d'exploitants agricoles mobilisés entreprises estoniennes emblématique Gatti chambre assure sur le les défis barrage de la paille, premières étape de la transformation du chanvre permettant la réalisation d'isolant d'enduits de béton et de blocs de chanvre comment dans ces conditions, explique les difficultés de mise en oeuvre des produits issus du chanvre dans le bâtiment, certes, la décision de l'Agence qualité construction qui avait rejeté l'an dernier les règles professionnelles édictées dans le but de massifier la construction en chambre est derrière nous et l'on doit se féliciter du soutien apporté aux nouvelles règles professionnelles dont la validation devrait intervenir prochainement, mais une autre entrave à l'usage du chanvre dans le bâtiment résulte de l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de valoriser financièrement le béton de chant, par le biais des certificats d'économie d'énergie, ce dispositif requiert en effet une certification sur les matériaux employés garanti par l'Association pour la certification des matériaux isolants, les règles professionnelles ne saurait tenir lieu de certification, or les performances thermiques remarquable chanvre ses capacités hydro-thermique inégalée, son pouvoir d'absorption des sons et sa résistance au feu sont amplement démontré un sujet d'inquiétude supplémentaire: tiens, au fait que la plupart des maîtres d'oeuvre sur des entreprises artisanales ou des PME spécialisées ne disposant pas toujours des moyens de financer la démarche de qualité permettant l'obtention du Label reconnu garant d'environnement, les maîtres d'Oeuvres ne peuvent donc pas prétendre aux aides de l'état aussi de la rénovation de l'habitat, enfin la filière manque singulièrement de moyens pour financer des fiches de déclarations environnementales et sanitaires nécessaires au respect de la nouvelle réglementation environnementale 2020 R E 2020, tous ces freins normatif ont une conséquence majeure : l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments n'est obtenu que par l'emploi de matériaux issus de grands groupes industriels dont l'impact environnemental et énergétique à la production et plus défavorable que pour les matériaux biosourcés alors que l'optimisation des ressources naturelles est indispensable pour assurer la transition énergétique et que la France peut se prévaloir d'être le leader européen de la production de chanvre, je souhaiterais que le gouvernement prenne des initiatives importantes pour obtenir la levée des contraintes pesant sur son utilisation dans le secteur de la construction, en particulier, il me paraît indispensable d'accompagner cette levée des restrictions par des mesures fiscales propres à soutenir le développement significatif des filières locales biosourcés dont celle du chanvre, permettez-moi de vous demander, Madame la Ministre, d'engager une concertation interministérielle sur ce sujet, mais c'est à ces conditions que notre pays pourra participer pleinement et rapidement à la transition énergétique rendue indispensable par la hausse exponentielle du prix de l'énergie dont souffrent nos concitoyens et des pans entiers de notre économie, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 4 minutes. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour commencer, je tiens à saluer les auteurs de cette proposition de résolution notamment notre collègue Guillaume Gontard et les membres du groupe écologiste solidarité et territoires, alors que le sujet de la filière chambre semble être récemment revenu sur le devant de la scène, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une culture très ancienne et qu'elle a connu une institut nia Lisa Sion en France dès 1932 avec la création de la Fédération nationale des producteurs de chambre grâce à la multiplicité de ses usages et de ses nombreuses vertus la filière chambre déjà un poids économique non négligeable et surtout des perspectives de développement particulièrement importante en effet en 2020 la filière chambre la filière française du chambre comptait plus de 1400 producteurs pour 17000 hectares exploités avec une surface de production multipliée par 3 en 15 ans. Grâce à ce dynamisme, la France est le 1er producteur européen de chambre et le 4ème mondial et pour une fois et je pense notamment, et c'est dommage, il est absent aujourd'hui aux auteurs du récent rapport sénatorial sur la compétitivité de la ferme France nous pouvons collectivement nous féliciter du dynamisme de cette filière malheureusement cette culture a toujours eu mauvaise presse, principalement à cause de la production de sa fleur aux effets psychotropes le cannabis avec les connaissances scientifiques et techniques que nous avons aujourd'hui, il convient de sortir des clichés de se rendre compte de la diversité des usages et des bénéfices du chambre en tant qu'agriculteur, je souhaite insister sur les opportunités agro-écologique de la production du chambre en effet cette dernière ne nécessite pas d'insecticide, pas de fongicides, pas d'herbicides et particulièrement économe en eau par la hauteur et la densité de cette plante, il est également un formidable réservoir à biodiversité qui peut pleinement s'inscrire dans l'indispensable rotation des cultures et dans l'entretien des sols, c'est donc une culture particulièrement saine qui peut être une puissante crise de vocation pour les jeunes agriculteurs qui ont la volonté de développer une agriculture plus vertueuses plus vertueux sur le plan environnemental et ainsi apporter une partie de la solution au problème du renouvellement des générations face aux difficultés économiques que rencontre de nombreux agriculteurs, le prix de revente de kilos de de fleurs CBD à environ 600 euros pour l'année 2022 peut également être une opportunité de développement pour le monde agricole bien sûr pour me permettre cela, et c'est l'objectif principal de cette résolution, il est nécessaire d'avoir une réglementation adaptée à la filière, notamment en permettant la vente de fleurs et de feuilles brutes et injuste, accompagnement par les pouvoirs publics, Swissair, dernier point je rejoins pleinement les recommandations de la proposition de la résolution tout particulièrement sur l'ouverture de la et cette filière à cette filière et l'obligation de déclaration des cultures pour être incompatibilité avec les obligations de la PAC, comme pour toutes les filières, la labellisation et la mise en conformité avec les critères permettront de réaliser un cadrage et ainsi d'éviter des dérives qui peuvent être facilement associé à cette culture. Enfin, et sur un plan économique plus globale, il est important de souligner que la diversité des usages du chambre lui permet d'avoir des perspectives de débouchés dans des filières très variés, mon collègue Gilbert Luc Domino's a justement abordé les secteurs du textile et du bâtiment, et nous pourrions également cité l'alimentation humaine, avec des graines particulièrement riche en protéines, l'alimentation animale avec les graines de chefs de Nice et bien sûr la filière papier avec près de 7 millions de consommateurs le CBD peut être une réelle opportunité pour les buralistes également, dont le nombre a diminué de 27 % en 20 ans et qui possède l'expertise et les compétences pour assurer la vente d'un tel produit ainsi, madame la ministre, alors que votre gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à soutenir le développement de la filière chambre, il est aujourd'hui essentiel d'apporter une clarification sur la réglementation autour du CBD, comme le prévoit l'alinéa 49, cette proposition de résolution, seul un appui aux acteurs de la filière et une précision sur le cadre légal et réglementaire permettront un développement et un développement, un réel développement de la filière française du chambre, mes chers collègues, en soulignant encore une fois la qualité de ses propositions de résolution et les différents objectifs mis en avant par ce texte, je vous invite à largement soutenir l'adoption de cette résolution comme nous le ferons au sein du groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, la parole est à madame la présidente Annie. Que Billon pour le groupe Union centriste et pour quatre minutes.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si aujourd'hui les voiles des monocoques du Vendée Globe ne sont pas constitués de fibres de chanvre, celle de la flotte de Louis XIV, la filière économique et du chanvre a ainsi connu ses heures de gloire au XVII et XVIIIe siècles avant de péricliter la confusion compréhensible entre le cannabis et la fleur de chambre ayant conduit à une marge une marginalisation de sa production à partir des années 90 émancipant complètement de l'ombre du cannabis, la filière renaît en s'appuyant sur des acteurs locaux, créateur d'emplois, nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution à l'issue d'initiative de nos collègues du groupe écologiste je salue cette initiative car elle nous permet de mettre en lumière, de belles entreprises dans nos territoires d'encourager une filière tout en ne donnant aucun signal en faveur de la légalisation de la dépénalisation du cannabis : agriculture, textile ou BTP la filière du chanvre sous ses différentes expressions a ainsi un véritable potentiel économique qu'il ne faut pas négliger cela fait ainsi plus de 20 ans que le secteur de la construction et du bâtiment s'appuie sur le chambre tant pour ses propriétés isolantes que pour la restauration d'habitation, je tiens à saluer, à ce titre la création il y a bientôt 25 ans, de l'association construire en chambre qui oeuvrent pour la valorisation de la filière depuis 2 décennies, c'est ainsi toute une économie qui s'est développée pour favoriser l'utilisation du chambre on s'appuyant sur ses qualités gros thermique sa durabilité et sa très bonne régulation de l'humidité, que cela soit, que cela soit là, je ne vote ou la fibre de chanvre cette plante a des débouchés économiques qu'il convient de valoriser en Vendée, cela fait plus de dix ans que la coopérative cava que je connais bien, a fait du chanvre un matériel essentiel dans le cadre de la construction bio-sourcés à l'heure où la rénovation énergétique des bâtiments est un pilier de la relance verte appelée de ses voeux par le gouvernement, il nous faut donner les moyens aux entreprises de la filière, les matériaux biosourcés doivent contribuer à la décarbonation de nos bâtiments, cette proposition de résolution pourrait à ce titre être utilement complété par 3 dispositifs l'élargissement de la formation des accompagnateurs rénovent au Mathieu Thériault bio-sourcés afin que les rénovations financée par l'outil ma priverait rénovant s'appuie également sur le chambre une meilleure valorisation de la capacité de stockage du carbone de du chanvre dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone 3 le lancement d'une réflexion au sujet de la mise en oeuvre d'un taux de TVA prenant mieux en compte les atouts des matériaux biosourcés pour conclure, l'adoption de cette proposition est un geste fort pour dire clairement notre soutien aux acteurs économiques de la filière : producteurs, coopératives industriels ainsi que l'ensemble des transformateurs, avec plus de 17000 hectares en France, il est temps de donner à la filière chambre un cadre légal stable permettant à l'activité de prospérer durablement et de se développer sainement, c'est pour cela qu'avec ma collègue daphné Ract-Madoux et l'ensemble du groupe Union centriste nous voterons en faveur de cette proposition issue du devront mesdames et messieurs les sénateurs. Merci, la parole est à monsieur Christian Klinger pour le groupe Les Républicains pour quatre minutes et vous essayez de pas tomber là dans l'escalier, ça va bien se passer.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, tout est bon dans le cochon, a-t-on coutume de dire : aujourd'hui j'ai envie de dire : tout est bon dans le chambre à la lecture de cette proposition de résolution au sortir d'un été marqué par la sécheresse et à l'heure des économies de chauffage le développement en France de la filière du chanvre plante sobre en haut et aux usages multiples paraît donc une évidence, c'est une plante qui pousse vite résistent à la sécheresse et qui enfin ne réclame pas d'apports en produits chimiques, les chiffres de la filière démontre l'intérêt de cette plante de moins de 4000 hectares en 1990 nous sommes passés à près de 22000 hectares en 2022 cultiver du chanvre, mais pourquoi faire tout, ou presque, si on en croit ses zélateurs Nat papier le chambre est encore utilisé pour produire des fibres textiles et permet aussi de fabriquer du papier sans abattre d'arbre est apparu également le béton de chanvre un matériaux de construction, bio-sourcés dont les propriétés isolantes en font aujourd'hui un précieux atout puis des fibres encore plus technique, notamment dans l'industrie automobile, sont devenus des alternatives aux fibres de verre beaucoup plus polluantes, les graines riches en protéines sont utilisables dans l'alimentation animale comme humaine, cette plante est donc au coeur de nombreuses innovations d'une forte demande sociale et d'opportunités économiques, j'ai relevé plus de 600 produits dérivés breveté dans le monde dont la moitié proviennent malheureusement toujours de Chine, d'autres pays ont bien compris l'intérêt de cette culture et ce sont d'ores et déjà saisi de cette chance de développement à titre d'exemple, lorsque les États-Unis ont décidé de soutenir la filière, ils sont passés de 9000 à 33000 hectares en un an, à notre tour, nous devons soutenir cette filière et créer un écosystème favorable avec des règles claires et surtout des patients non, le débat autour du caractère psychotrope du cannabis fibre graines la plante, vous le savez, a aussi des feuilles et des fleurs, se pose alors un problème de réglementation au sujet du chanvre, bien-être, laquelle paraît à ce jour, assez confuses autorisé par l'Europe, la commercialisation des fleurs et feuilles a été suspendu par un arrêté, lequel a été invalidé par le Conseil d'État en janvier dernier, la Cour de cassation, quant à elle, a légalisé la commercialisation de ces produits, bref, si nous voulons une filière française d'excellence, celle des extraits de chambre, il s'agit de donner à nos entreprises la possibilité d'investir sereinement et pleinement ses marchés d'avenir en clarifiant les réglementations applicables aux différents produits finis et en les alignant sur celle de nos homologues européens et britanniques pour jouer à armes égales, le chanvre, une croissance très simple, depuis l'implantation jusqu'à la récolte, cette dernière nécessite un matériel spécifique et un temps d'intervention plus long que la majorité des cultures, la graine étant fragile et la paille demandant plusieurs interventions avant sa transformation, la culture de chambre nécessite donc des outils spécialisés et donc des investissements, or les investissements demeureront frileux, tant que les règles ne sont pas clairs ni pérenne la position de la France, elle reste figé reviendra donc à Val à favoriser les nos pays voisins, sans aucune justification rationnelle, il y a un an, nous avions eu un débat ici même sur ce sujet, le gouvernement a annoncé sa volonté, je cite, de mettre en place un cadre réglementaire pour permettre le développement sécurisé de la filière, force est de constater que le dossier n'a pas bougé mais pourquoi attendre la loi de transition énergétique demande de concevoir des bâtiments à énergie positive, faisons en sorte que ces matériaux de construction biosourcés soit sur notre marché, mes chers collègues, vous l'aurez donc compris si tout est bon dans le cochon, c'est le cas du chanvre, aussi, je vous remercie. Si chaque fois. Si, si. La parole est à Madame Dominique Faure, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Merci madame la présidente, monsieur le président de la commission. Mesdames et messieurs les sénateurs, je dois reconnaître au groupe écologiste solidarité territoires et à son président Guillaume Gontard une constance qui l'honore, puisque le sénat avait initié ce débat important sur l'avenir de la filière du chanvre en février dernier à votre initiative, cette proposition de résolution va nous permettre d'approfondir les échanges que vous aviez alors eu avec le gouvernement et montres par la diversité des soutiens qu'elle a recueillis sur ces bancs, toute l'importance de ce sujet ainsi que sa complexité, cela a été dit, il s'agit, je crois, d'un point de consensus, mais je me permets de souligner à nouveau le chanvre est une filière dont nous devons soutenir le développement en raison des opportunités qu'elle offre, d'un point de vue agro-écologique, il s'agit en effet d'une culture qui nécessitent une quantité relativement limitée d'azote pas irrigation or conditions climatiques exceptionnelles du fait de ses racines profondes, elle ne nécessite aucun traitement phytosanitaire, ce qui lui fait également de la biomasse produite un réservoir de biodiversité d'insectes et d'anthropologues, dont notamment des espèces régulatrice des ravageurs de cultures en outre le chambre participe à l'allongement des rotations des exploitations de grandes cultures et à la diversité des à seulement enfin l'utilisation de plus en plus répandue de ces produits dans le bâtiment en fait un produit agricole contribuant à stocker du carbone au lieu d'en émettre cela sera important de veiller à ce que l'amont agricole soit bien considérés dans le calcul des crédits carbone générées, l'enjeu est que les producteurs soient équitablement rémunérés par la vente de ces crédits carbone ce qui participera à l'attractivité de la culture du Champ pour nos agriculteurs, nous veillerons donc est-ce que cela soit bien pris en compte. Par le comité scientifique et technique du Label bas-carbone dans les méthodologies de calcul pour le chambre pour le chanvre et plus gros globalement pour les biomasse agricole valorisé dans les autres secteurs industriels,

Fesneau. Significativement en faveur du développement de la filière au ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire à travers le dialogue constant qu'il entretient avec Inter chambre l'inter-profession mais aussi financièrement, outre les aides classiques de la politique agricole commune, la filière chambre bénéficient d'une aide couplée quatre-vingt-seize euros à l'hectare, si la production et contractualiser. Et que la variété et certifiée. En tout cas, les enjeux sont majeurs pour la France 1er producteur de chambre au niveau européen mais aussi mondial, le développement de la filière chanvre n'est d'ailleurs pas uniquement un objectif que nous devons nous fixer en matière agricole et alimentaire puisque les débouchés qu'elles offrent peuvent constituer des atouts intéressants pour notre pays en matière énergétique écologique ou industrielle Je vais juste interrompre 2 secondes excusez moi sincèrement, je vais vous demander quand même un peu de respect et de parler tous un peu plus bas ou de d'écouter madame la ministre a je vous remercie. Dans un contexte d'accroissement des surfaces qui ont été multipliées par 3 en 10 ans, la culture du chanvre alimente ainsi de nombreux marchés qui vont de la papeterie à l'automobile, du bâtiment au jardinage, en passant par la plasturgie, l'alimentation animale et humaine, ou encore le textile, j'ajoute : il s'agit d'un point qui me semble absolument essentiel du point de vue du dynamisme et de la vitalité économique de nos territoires, notamment ruraux que la filière se caractérise notamment par l'existence d'un grand nombre d'acteurs de taille modeste fonctionnant en circuit court avec un ancrage territorial particulièrement fort, j'y suis, comme vous, profondément attaché, la proposition de résolution examiné aujourd'hui s'inscrit résolument dans cette logique de soutien au développement de la filière chambre en France et le gouvernement estime que cette initiative sénatoriale. Viendra utilement enrichir les réflexions à mener dans cette perspective, le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire est prêt à continuer à travailler en lien très étroit avec le Sénat sur cette dimension agricole du sujet, j'en viens maintenant au second volet de cette proposition de résolution qui concerne un sujet qui dépasse largement le Champ de l'agriculture, celui de l'amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre, il s'agit d'un sujet auquel le gouvernement apporte une attention toute particulière, et sur lequel, loin des caricatures qui peuvent parfois caractérisé ces débats, ce n'est pas ici le cas, bien sûr, nous souhaitons poser les enjeux avec exigence et méthodes, je voudrais en 1er lieu aller dans le sens de ce qui a été dit par plusieurs orateurs, oui il existe incontestablement des enjeux autour de la réglementation des produits issus du chanvre, dont la consommation de cannabidiol mais donc il existe incontestablement des enjeux autour de cette réglementation des produits issus du Champ et naturellement le plus évident, mais pas le seul ces sujets importants ont été posées avec plus d'acuité encore avec la suspension par le Conseil d'État du cadre réglementaire global, dont la France s'était dotée, devrait devait permettre le développement sécurisé de la filière agricole du Champ, ainsi que des activités économiques liées à la production d'extraits de chambre à la commercialisation de produits qui les intègrent tout en garantissant la protection des consommatrices et des consommateurs et le maintien de la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, l'absence d'une réglementation claire sous la ville est vrai, un certain nombre de difficultés et, plus spécifiquement, j'en citerai trois une forme d'instabilité pour les acteurs de la filière, que ce soit le monde agricole, industriel, les laboratoires ou le commerce de détail qui manque de visibilité dans la conduite de leur projet économique, deuxièmement une commercialisation possible en France, mais avec une immense majorité de fleurs et d'extraits commercialisé issus de l'importation, ce qui est un enjeu pour notre filière pour notre filière troisièmement, un sujet de sécurité en termes de consommation car je tiens à le souligner ici, si le cannabidiol n'est pas classé comme un stupéfiant, il s'agit tout de même une substance à effet psycho actifs dont les risques pour la santé sont encore en cours d'expertise partant de ces constats, je voudrais partager avec vous quelques éléments de réflexion en 1er lieu que nous dit le Conseil d'État que les produits dont la teneur en tétrahydrocannabinol, THC n'est pas supérieur à 0 3 pour 100 ne revêtent pas un degré de nocivité pour la santé, justifiant une mesure d'interdiction générale et absolue de leurs ventes et de leur consommation, en effet, il n'est pas,

c'est la raison pour laquelle je nous invite collectivement à la prudence sur ce sujet, mais aussi au travail scientifique que mène actuellement l'Autorité européenne de sécurité des aliments car il nous semble que seule la science doit éclairer nos décisions, s'agissant d'un sujet aussi délicat, il s'agit je crois du chemin que nous devons emprunter sans précipitation, deuxièmement, je tiens à souligner qu'en l'état actuel de la réglementation, les services de police et de gendarmerie seront recherchées relever des infractions comme la provocation, même non suivies d'effet à l'usage illicite de stupéfiants, il n'est pas acceptable par exemple que des publicités en faveur du cannabidiol entretiennent la confusion avec le cannabis et font ainsi indirectement la promotion de ce stupéfiant, en dépit de la suspension de certaines dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2021, nous ne sommes donc pas dans un no man s'land juridique, s'agissant de ce sujet et nous sommes bel et bien en mesure de lutter contre tout ce qui peut s'apparenter à la promotion et à la banalisation du cannabis, il s'agit, je le rappelle, de la manière la plus claire possible de la position ferme et constante du gouvernement sur ces sujets, au-delà de ces réponses qui sont absolument nécessaires, des réflexions inter ministériels sont en cours sur ce qui pourrait constituer une politique de contrôle aboutit sur la commercialisation des extraits de chanvre certaines des orientations de cette proposition de résolution pourrait d'ailleurs en partie s'intégrer dans le cadre de ses réflexions, je vois 3 enjeux à ces contrôles qui relèvent de la compétence à la fois de, de, de nos services et des services de la DGCCRF, le premier de contrôler l'absence de pratique commerciale trompeuse et de tromperie sur les qualités substantielles du produit relevant du code de la consommation, notamment en cas d'allégations trompeuses et notamment d'allégations de santé non autorisées ou thérapeutiques en lien avec l'utilisation d'extraits de chant le 2ème enjeu de donner des informations claires aux consommateurs sur les bonnes pratiques d'utilisation et et les publics pour lesquels la consommation d'extraits de champs est à éviter, jeunes enfants, femmes enceintes, enfin il y a un enjeu à réaliser des contrôles aléatoires sur les produits commercialisés en France afin de vérifier notamment l'absence de contamination des extraits par le THC et éviter ainsi des risques de santé publique, ces produits n'échapperont pas au retrait et rappel en cas de non-conformité, j'ajoute, s'agissant du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire que nouveau conseil scientifique piloté par l'interprofession Inter chambre a été créé en février 2022 afin d'accompagner au mieux les agriculteurs qui souhaitent produire les fleurs de chanvre, 3 groupes de travail ont été constitués sur la génétique sur l'itinéraire technique du chambre à destination de la production de fleurs sur la mécanisation de la récolte des fleurs, une feuille de route est donc en en cours de définition, enfin, je tiens tout de même. à vous faire partager des interrogations sur les conséquences agricole, alimentaire et environnementale que pourrait avoir un développement débridé des débouchés liés à la consommation de cannabidiol et autres extrait extrait de chant qui se vendent à prix d'or, allons-nous nous nourrir d'extraits de chambre à ce jour, la production de chambre à fleurs et bien distinctes. De celle du chanvre destiné à la production de graines et de fibres, il nous appartient ainsi de peser les conséquences d'un tel choix sur les autres débouchés qui pourrait mécaniquement perdre de leur attractivité parfois déjà déjà fragiles, je pense en particulier à l'alimentation humaine et animale, qui est un enjeu de souveraineté alimentaire ou encore à l'isolation des bâtiments en jeu d'indépendance énergétique et de transition écologique, or ce sont bien ses priorités qui sont à l'agenda des priorités du gouvernement, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les sénateurs, sans en partager la totalité des orientations en particulier s'agissant des préconisations formulées sur la réglementation des produits issus du Champ le gouvernement considère que cette proposition de résolution et très utile au débat et se saisira du vote au Sénat pour poursuivre et accélérer les réflexions indispensable un développement mais. Et ambitieux de la filière, je vous remercie. Alors, nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution la conférence déprécie des présidents a décidé que les interventions des orateurs, explications de vote, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste sur la proposition de résolution, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 dur règlement le scrutin est ouvert.

OK, plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos.

voici le résultat du scrutin numéro 55 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence, nombre de votants 208 Nombre de suffrages exprimés 186 pour l'adoption 179 contre cette, le Sénat a adopté. Je vais suspendre la séance vraiment. Quelques instants pour permettre à chacun de s'installer pour l'examen du prochain point à l'ordre du jour, la séance est suspendue.

La séance est reprise, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Alors je vais donner la parole à Madame Frédérique Puissat, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire pour cinq minutes et je vais demander que les discussions se passent dans le couloir, merci beaucoup, merci, cher collègue. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales chères Catherine, mes chers collègues. La commission mixte paritaire, réunie le 9 novembre dernier est parvenu à un accord sur le projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, un texte auquel le Sénat s'est attaché à donner du sens au delà d'une prorogation des règles actuelles du régime d'assurance chômage, avec mon collègue rapporteur Olivier et non que je salue, je tiens à saluer Marc Ferracci, rapporteur pour l'Assemblée nationale, avec qui les échanges en amont de la CMU CMP ont été nourris et empreint de sincérité mais aussi de beaucoup d'exigence, remets reviendrait ici que sur les points les plus saillants du texte qui vous est proposé d'adopter aujourd'hui à l'article 1er qui a constitué un point central des discussions, la CMP a adopté une rédaction de compromis qui répond à la volonté du Sénat de restaurer la place des partenaires sociaux dans la définition des règles de l'assurance chômage, comme le prévoyait le texte initial, le gouvernement sera autorisé à prendre par décret en Conseil d'État, les mesures d'application du régime d'assurance chômage, jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi qu'à prolonger l'application du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage, jusqu'au 31 août 2024 en revanche la rédaction issu de la CMP conserve l'apport du Sénat prévoyant que le gouvernement devra engager conformément à l'article L-1 du code du travail, une concertation avec les partenaires sociaux sur la gouvernance de l'assurance chômage, mais aussi sur les conditions de l'équilibre financier du régime qui pourra déboucher sur une négociation, le document d'orientation invitera notamment les partenaires sociaux à négocier sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage issues de la réforme de 2018 et que le Sénat avait entendu supprimer l'inscription par le Sénat dans la loi du principe de contrat cyclicité que le gouvernement entendait mettre en neuf, par décret, a été maintenu par la CMP, par ailleurs, afin de revenir à la vocation première de l'assurance chômage d'indemniser la privation involontaire d'emploi Le Sénat avait introduit 2 articles visant à supprimer l'allocation en cas de refus de CDI, la CMP a pris en compte le risque juridique que comporter la différence de traitement entre différentes catégories de salariés, et a donc adopté à l'article 1er bis à à une rédaction de compromis concernant à la fois les fins de CDD et les fins de mission d'intérim dans les 2 cas, l'indemnisation du chômage sera supprimée après 2 refus de CDI sur un emploi similaire, elle a également renvoyé les modalités d'application du dispositif à un décret en Conseil d'État et clarifier son articulation avec le PPA, nous pouvons nous féliciter que le Sénat était entendu sur ce point, ne pouvons en revanche nous sommes particulièrement attentifs, madame la Ministre, à ce que son application ne donne ne donne pas lieu comme j'ai pu le lire dans la presse régulièrement à une usine à gaz, mais bien des solutions opérationnelles permettant une mise en oeuvre effective de cette mesure, la balle madame la Ministre est clairement dans votre camp dorénavant à l'article de le Sénat avait proposé des évolutions substantielles du bonus-malus sur les contributions d'assurance chômage, la CMP, revenu à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui apporte une transparence bienvenue aux employeurs concernés il conviendra toutefois après 2 ans d'application du dispositif de tirer les conséquences qui s'imposent, il s'avère inadapté à l'article IV concernant la VAE, le Sénat avait souhaité sortir d'une approche par statut en posant le principe d'une VAE ouverte à toute personne dont l'expérience est en lien avec la certification disait la CMP a conservé cet apport qui doit contribuer à donner un nouveau souffle à cette voie d'obtention d'une certification, elle a également maintenu la précision selon laquelle l'émission du GIP nationale créée par le projet de loi pour mettre en oeuvre les services publics, de la VAE de devrait être assuré en tenant compte des besoins de qualification selon les territoires, en revanche, la CMP sur la joue, par le Sénat de 2 membres de droit supplémentaire au sein du GIP et sur le principe de sa présidence par un président du conseil régional c'est précisant pour être défini dans le cas de la de la convention constitue, site du give du GIP, sans que la loi fiche excessivement sa gouvernance, mon collègue Olivier Henno, qui a travaillé ce point on parlera bien mieux que moi, tout à l'heure au total ce texte reflète notre ambition de redonner une chance au paritarisme et notre préoccupation d'adapter les règles d'indemnisation du chômage aux réalités actuelles du marché du travail au nom de la commission il paritaire, je vous propose donc de l'adopter et je profite de cette intervention pour remercier les administrateurs du Sénat messieurs luzerne Asia vie ainsi que Madame Delphine Mancel et t'adresser un petit clin d'oeil à mon fidèle compagnon dans ce texte, Olivier et non merci beaucoup. Merci beaucoup, la parole est à Madame Carole Grandjean. Jean Ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci madame la présidente, madame la présidente de commission madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je tiens en 1er lieu à excuser Olivier Dussopt, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, je me réjouis néanmoins de de l'accord trouvé entre votre chambre et celle des députés en commission mixte paritaire, cet accord s'explique, je crois, notamment par la qualité des débats pendant tout l'examen de ce projet de loi, je tiens à remercier l'ensemble des parlementaires qui ont oeuvré à rendre possible un compromis au profit de l'intérêt général, l'esprit de responsabilité et le sens de l'intérêt général, ont permis de parvenir à un texte à la fois équilibré et à la hauteur des enjeux qui marque une étape supplémentaire vers le plein emploi, je veux également saluer également le travail exigeant des 2 rapporteurs madame Frédérique Puissat et monsieur Olivier Henno, vous avez, par voie d'amendement apporté de nombreuses modifications importantes au texte et je crois que nous pouvons vous en remercier collectivement par ce texte, hein, nous préservons les droits des demandeurs d'emploi, il confère au gouvernement la possibilité de prolonger les droits d'indemnisation pour 14 mois jusqu'au 31 décembre décembre 2023 il prolonge également le bonus malus, jusqu'au 31 2022 31 déc 2024 ce dispositif nous permet d'encourager les entreprises à moins recourir aux contrats de très longue durée, par ailleurs, à la faveur d'un amendement proposé par votre chambre, le texte issu de la commission mixte paritaire prévoira explicitement la possibilité de faire varier les règles de l'assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail, cet amendement est non seulement utile à en terme de lisibilité, mais il témoigne également de la volonté commune des législateurs de sécuriser de soutenir et d'encourager l'arrêt. Forme que nous sommes en train de mener, en concertation avec les partenaires sociaux à ce titre, Olivier Dussopt réunira les partenaires sociaux le 21 novembre prochain afin de conclure les concertations que nous avons conduite depuis le 17 octobre dernier la solution que nous retiendrons qui sera juste et équilibré, s'appuiera sur une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi au regard des opportunités des opportunités sur le marché du travail cette modulation, elle viendra soutenir notre activité économique à un moment où nous avons, nous en avons considérablement besoin ou à titre d'exemple, 30 pour 100 des entreprises renoncent à une partie de leur activité, pour des raisons de pénurie de main-d'oeuvre, contrairement à ce que nous avons pu entendre cette réforme ne pénalisera pas les demandeurs d'emploi les plus fragiles, ainsi la réforme ne reviendra pas sur les conditions d'affiliation minimale: elle ne diminuera donc pas le nombre de personnes s'ouvrant des droits à l'assurance chômage, vous avez également apporter une clarification législative sur l'abandon de poste désormais l'abandon de poste prévaut prévaudra présomption et je veux bien souligner ici, il s'agit bien d'une présomption de démission, la nuance est importante, je veux m'y arrêter quelques secondes cette disposition sera tout d'abord, suivi d'un décret, l'abandon de poste n'étant pas vraiment formalisé par le code du travail, elle aboutissait à une situation de faute grave or il n'est pas anodin d'être licencié pour faute grave et ce processus et la possibilité de toucher des indemnités de licenciement, la nouvelle procédure qui verrait le jour en cas d'adoption permettrait d'expliciter les véritables causes sous-jacentes à l'abandon de poste la démission s'imposera lorsque le salarié arrête d'exécuter son contrat de travail sans prévenir une procédure de mise en demeure par l'employeur est prévu, ce qui permettrait d'écarter la démission lorsque l'abandon de poste justifie par des motifs de santé ou de sécurité par exemple, prenons également acte de la volonté des législateurs d'encadrer les refus de proposition d'embauche des du en CDI qui font suite à des contrats d'intérim ou de contrat à durée les ajustements et encadrement nécessaire proposé en commission mixte paritaire et l'investissement transparaissent disant sur ce sujet ont permis d'aboutir à un compromis, vous avez ainsi pris soin de préciser que les CDI refuser doivent être conformes au profil de l'offre raisonnable d'emploi telle que précisée par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi, cette précision apparaît nécessaire afin de ne pas risquer de réduire la part de demandeurs d'emploi qui acceptent d'occuper un emploi en attente de trouver un emploi plus conforme à leur projet professionnel, cette disposition a également permis d'ouvrir un débat intéressant sur les conditions d'attractivité et de fidélisation à certains métiers, ainsi que sur les nouveaux comportements sur le marché du travail, notamment celui des jeunes, enfin vous avez souhaité intégrer les centres de gestion de la fonction publique territoriale dans le processus d'accès à l'assurance chômage des agents des collectivités territoriales, démissionnaire, et qui, dans la suite de leur trajectoire se retrouvent en situation de percevoir l'assurance chômage, selon la réglementation de l'assurance chômage, dans certains cas, les collectivités locales se retrouvent en situation de devoir payer le montant des allocations versées nous sommes sensibles à cette curiosité du droit qui peut parfois mettre dans la difficulté financières certaines collectivités locales, et donc effectivement ces évolutions ont trouvé place dans ce texte, cette nouvelle disposition ne suffira probablement pas totalement et Olivier Dussopt là effectivement indiqué devant votre chambre, il s'est engagé à examiner ce sujet avec mes collègues ministres de la fonction publique et des collectivités locales afin de trouver une solution définitive, vous avez également confirmé la volonté parlementaire forte de refonder un dispositif de validation des acquis de l'expérience, plus moderne, plus simple, plus sécurisant pour ses candidats en offrant un nouveau cadre de coopération autour de la validation des acquis de l'expérience réussiront ainsi à concilier, j'ai été sensible des objectifs nationaux et des stratégies locales de développement des emplois et des compétences, ce texte fonde un nouveau service public pour notre pays, celui d'une reconnaissance élargie des compétences des actifs dans une véritable logique d'universalité que la majorité sénatoriale a porté et promu tout au long des débats, c'est donc une validation des acquis d'expérience dont nous aurons ouvert grand les portes et que nous sommes fiers de porter aujourd'hui devant vous, les avancées permises par ce projet de loi sont nombreuses, elles sont importantes, elles constituent des jalons sur le chemin du plein emploi, aux côtés d'autres leviers que nous souhaitons mettre en oeuvre cette réforme est une première réalisation dont nous pouvons collectivement nous féliciter, vous l'aurez compris le gouvernement était évidemment favorable à l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire, je vous remercie, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale, le texte élaboré par la commission mixte. Paris-se prononce par un seul vote sur l'ensemble de ce texte, en ne retenant que les amendements présentés ou accepté par le gouvernement, en conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservée,

Merci, il avait du gouvernement merci. Et de l'amendement numéro 2 un amendement de coordination merci avec du gouvernement favorable, merci beaucoup, alors nous passons donc aux explications de vote des groupes à raison d'un orateur par groupe,

mais pas rapporteur spécial, mais on se retrouvera comme rapporteurs spéciaux tout à l'heure, tout à l'heure, mes chers collègues, atteindre le plein emploi, c'est évidemment un objectif économique, le plein emploi, c'est plus de ressources et moins de dépenses, c'est la formule la plus simple pour équilibrer le régime sans diminuer le montant des allocations. Mais atteindre le plein emploi, c'est un objectif surtout sociale, d'abord parce que pour trouver sa place dans la société, mieux vaut un travail que des allocations, ensuite parce que, lorsque le marché du travail tendu le pouvoir de négociation des travailleurs augmente, c'est un fait, notre groupe soutient la politique du gouvernement pour atteindre cet objectif, la réforme de l'assurance-chômage en constitue évidemment un axe incontournable pour atteindre cet objectif, il faudra aussi réformer les retraites ajuster la politique en faveur de l'apprentissage, développer l'enseignement supérieur professionnel pardon recadrer la formation continue, tout cela fait partie de l'agenda du gouvernement et ne seront en soutien de ces réformes, mais la priorité était bien de réformer l'assurance chômage, d'abord pour des raisons de calendrier, les règles encore en vigueur, devait être prolongée, la majorité sénatoriale souhaitait anticiper le retour aux parents de charisme, de gestion, je crois qu'il vaut mieux laisser davantage de temps aux partenaires sociaux pour définir les prochaines règles c'est pourquoi la prolongation des règles actuelles jusqu'au 31 décembre 2023 dans le va dans cela donne de la visibilité tant pour les partenaires sociaux que pour les demandeurs d'emploi, cela permet aussi d'anticiper les nouvelles modalités de négociation prévues par le texte, à cet égard la version issue de la commission mixte paritaire est clair : les partenaires sociaux devront chercher à équilibrer les finances du régime, c'était un amendement de précision que nous portions au Sénat je me me réjouis qu'il figure bien dans la loi. Certains points du texte ont provoqué quelques interrogations. Je pense notamment à la présomption d'émission pour les abandons de poste sur ce sujet, personnellement, je comprends la logique de la mesure, mais je doute. De son effet réel sur le marché du travail, à titre personnel, je dois avouer que je crains qu'il ne fasse peser sur les PME des risques contentieux plus important qu'avant, et les propos de Madame la Ministre, sur le distinguo entre la démission présumé ah bon santé pas santé harcèlement moral évidemment nécessairement aussi enfin toutes les exceptions, me font craindre que, au final, en partant d'une bonne idée, ce soit les PME qui n'ont pas de services de ressources humaines qui qui

le compromis issu de la CMP me semble plutôt modérée, j'espère qu'il suffira pour atténuer ce phénomène, c'est un phénomène qui désespère autant les chefs d'entreprises qui veulent recruter de façon pérenne que les demandeurs d'emploi qui cherche un CDI, cela a été dit et répété par la par la rapporteur pour le Sénat, notre collègue Frédérick puis à l'assurance chômage doit rester un filet de sécurité pour les salariés involontairement privés d'emploi, nous soutenons cette ligne de bon sens concernant la contrat cyclicité des règles d'assurance chômage et l'application du bonus-malus, c'est au gouvernement d'agir, nous espérons qu'il suivra cette ligne avec un objectif clair : garantir l'équilibre financier du régime et engagé le désir d'endettement de l'Unédic, vous l'aurez compris le groupe les indépendants

Merci madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, avec l'amendement retraites votée récemment ce projet néolibéral relatifs au fonctionnement du marché du travail marque un nouveau recul pour les droits des travailleurs il pervertit le système assurantiel en le mettant au service, non de la protection du risque, suite à un dissentiment mais d'une politique de baisse des allocations pour affaiblir la capacité des demandeurs d'emploi de négocier des conditions d'emploi digne ah si des dispositions qui ont été introduites ici est validée par la CMP, comme la suppression des allocations après 2 refus de CDI suite à des CDD qui en plus d'être une usine à gaz perpétue la politique du soupçon et de la menace envers les chômeurs, accusé de préférer les prestations de chômage au travail travail par lequel on feint de l'oublier, ils ont acquis ces droits opposé prestation et travail est un non-sens, mais je vous accorde que cette petite musique de division répété à satiété par les médias, fini par pénétrer les esprits, la majorité sénatoriale, bien sûr, mais après d'autres malheureusement. à la faveur d'un effet de loupe d'une extrême minorité de cas oh justifier un durcissement des modalités d'accès à l'assurance chômage, une diminution des allocations ou de la durée ayant pour effet et disons-le pour objet de réduire les marges de manoeuvre et d'arbitrage des demandeurs d'emploi pour les contraindre à accepter plus vite des employes de piètre qualité. c'est vérifié au Canada, pays qui sert de modèle ou les études ont montré que la contrainte cyclicité et le durcissement de l'accès à l'assurance chômage conduit les chômeurs à accepter des emplois moins rémunérés bloquant durablement leurs perspectives d'évolution de carrière, voilà l'objectif avec la baisse des dépenses, le texte offre un blanc-seing au gouvernement, désormais libre de moduler les règles de l'assurance chômage après un simulacre de concertation avec les partenaires sociaux privés de négociation car unanimement opposée à l'introduction de la cyclicité il faut avancer vite dans la libération du marché du travail. Et la reprise des droits des travailleurs tout à son objectif de plein emploi apparent à 5 % le gouvernement ignore les faits et la recherche, il refuse de questionner les causes réelles des tensions dans certains secteurs a, répétons-le, seulement 6 % des 3 millions d'offres déposées à Pôle emploi étaient non pourvus en 2021 soit 186000 emplois. selon Pôle emploi, les 3 quarts des recruteurs d'une offre non pourvues, reconnaissent que les conditions de travail du poste proposé peuvent décourager le candidat. Et l'adresse soulignait que les difficultés d'embauche dans certains secteurs en tension était lié aux conditions de travail dégradées et aux salaires insuffisants les offres non pourvues ont donc avoir essentiellement avec la non qualité de l'offre, ce qui explique selon les l'OFCE 60 % des chômeurs non indemnisés n'accepte pas plus ses employes la réforme aggravera la situation de précarité de beaucoup de chômeurs car non les allocations chômage ne des incite pas au travail et non, on ne gagne pas plus au chômage qu'en activité, selon l'Unédic, en moyenne, les personnes indemnisées au titre de l'assurance chômage perçoivent une allocation inférieure au seuil de pauvreté, 7 chômeurs indemnisés sur 10 reçoivent une allocation durant moins d'un an, près de la moitié des bénéficiaires de la queue de l'allocation chômage travaille déjà partiellement et selon l'adresse, il y a entre 25 et 42 % de non recours pour eux comme pour les 2 millions de personnes qui grossissent chaque année les rendu à long de chômage, cette réforme ne propose rien, mais grave en somme en ramenant le chômage à des aléas Moreau à des comportements individuels calculateur la petite semaine, vous refusez de questionner les causes structurelles qui relèvent de la dégradation des salaires et des conditions de travail comme de la perte de sens de beaucoup d'emplois, comme le souligne le sociologue Charles Wright Mills lorsque dans une nation plusieurs millions de salariés sont au chômage, on a affaire à un enjeu collectif l'énoncé correct du problème réclame l'examens préalables la site des institutions économico-politique de la société et non plus des seuls caractères propres aux individus, ce projet de loi aurait pu servir la cause du travail et des droits des travailleurs, il a choisi d'endosser le raisonnement partial et intéressé du patronat qui se l'amour sera ensuite de la non-motivation des travailleurs que vous réformes auront poussé à accepter des emplois non attractif, comme au Canada, elle ne résoudra pas la crise de l'attractivité et nous voterons le groupe écologiste contre merci. Mais merci, la parole est à monsieur Martin lévrier. Pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, ce n'était pas inéluctable ce mois-ci encore le taux de chômage a reculé de 0 1 point au sens du BIT se chiffrent corroborent la création de 84000 emplois dans le secteur privé au 3ème trimestre concrètement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, à l'Élysée, le taux de chômage est passé de près de 10 % à 7,3 ces résultats sont le fruit des actions menées par les gouvernements qui se sont succédé depuis 2017 et démontre que le plein emploi n'est pas une utopie, initialement composé de 5 articles, le texte s'est enrichi de 10 articles au cours de la navette parlementaire, parmi lesquels 2 ont été adoptés conformes 13 articles restait donc en discussion lors de la commission mixte paritaire du 9 novembre 2022, excusez-moi le chemin vers l'accord en CMP n'était pas tout tracé le compromis trouvé témoigne de la volonté des rapporteurs chargés de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d'agir en commun pour aller vers le plein emploi, je tiens à saluer le travail accompli par Madame la sénatrice, Frédérique Puissat, monsieur le sénateur, Olivier Henno et le député Marc Ferracci, à l'Assemblée nationale. Notre route est droite et la pente s'adoucit l'accord trouvé en commission mixte paritaire, tout en gardant les grands principes du texte initial, je pense notamment à la modulation des indemnités ou encore au rétablissement de la base légale relatives aux conditions pour être électeurs aux élections professionnelles, reprend les apports du Sénat sur la gouvernance de l'assurance chômage, les incitations à accepter un CDI dans un contexte de forte tension sur le marché du travail et sur les et sur la validation des acquis de l'expérience, la commission mixte paritaire a ainsi acté de l'ouverture d'une négociation interprofessionnelle sur la gouvernance de l'assurance chômage qui portera notamment sur l'équilibre financier du régime et l'opportunité de maintenir le document de cadrage de la suppression de l'allocation chômage après 2 refus de CDI à l'issue de contrats à durée déterminée ou de missions d'intérim, il tient compte du risque juridique que comportait la différence de traitement entre salariés en CDD et intérimaires, en revanche, si je me réjouis que la réforme de 2000 19 et permis de réduire la part de contrats courts dans les offres d'emploi disponibles, je concède ne pas être convaincu par ce durcissement des règles et pour cause, il tend à stigmatiser les personnes qui n'accepteraient pas un contrat à durée indéterminée et laissent à penser que seul ce type de contrat garantit la sécurité de l'emploi, pourtant, force est de constater que plus de la moitié des CDI sont rompues sous 2 ans, preuve que la flexibilité gagnant gagnant et plus efficace que la stigmatisation, enfin, la CMP a acté le principe de l'ouverture de la VAE à toute personne dont l'expérience est en lien avec la certification visée : les proches aidants pour le médico-social, bien évidemment, mais pas seulement les bénévoles trop entre autres patrons pour valoriser leurs expériences dans les associations, en promouvant la VAE au rang de voies de formation à part entière, l'article 4 du projet de loi considérablement enrichi par le gouvernement et les parlementaires vient concrétiser la crique à la création d'un véritable service public de la formation, rappelons que cette réforme a pour ambition d'atteindre l'objectif de 100000 VAE chaque année contre 30000 actuellement, vous l'aurez compris notre groupe se réjouit de que de l'Accord trouvé en CMP et votera ces conclusions issues d'un Beckham et équilibrée, qui évite un blocage de débat entre nos assemblées, ce texte répond à la pénurie de main-d'oeuvre en augmentant le nombre de personnes aptes à occuper un métier en tension et en accompagnant les revers les reconversions professionnelles des salariés, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Monique Lubin, pour le groupe socialiste, écologiste. Les républicains pour cinq minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission des affaires sociales, l'examen du projet de loi aura été l'occasion pour le gouvernement de montrer son vrai visage, il n'est plus dans le en même temps, mais confirme qu'il n'est ni de gauche ni de gauche, le groupe socialiste, écologiste et républicain n'était déjà pas d'accord avec l'évolution de l'assurance chômage, résultant de la réforme de 2018, c'est peu de dire que nous sommes aujourd'hui opposés à la radicalisation de ces dispositions et au sort dévolu aux partenaires sociaux ce texte qui, d'emblée, tourner le dos au paritarisme et dégrader les droits des travailleurs actée dès le début la contrat cyclicité qui serait inscrite dans le code du travail, elle a pourtant été un désastre dans les pays qui l'ont pratiquée comme c'est le cas au Canada, au vu de l'expérience de ce pays, l'instabilité que promet aux travailleurs cette disposition et l'arbitraire qui l'ouvre à leur détriment et pour nous tous une promesse de difficultés accrues dans de brefs délais, ce texte, déjà peu enthousiasmant est arrivée au Sénat encore durci par les débats de l'Assemblée nationale, les apports de la chambre basse aboutissent notamment à considéré comme démissionnaire tout salarié présumé fautif d'un abandon de poste et ainsi à le priver de toute indemnisation au titre du chômage cela atteste du choix de gouverner aux préjugés un incriminant le travailleur aucune donnée objective, a fortiori chiffrée n'est avancée pour étayer une telle mesure ne serait-ce que par les rapporteurs avec cette mesure, nous risquons de compliquer la mise au jour des raisons pour lesquelles l'abandon de poste, il y aura eu raison potentiellement liées aux caractéristiques inhérentes au management de l'organisation que le travailleur, c'est résolu de quitter aux conditions de travail qui lui sont imposées de maigre protection ont certes été rajouté dans le texte, mais elles sont très insuffisantes, le fêter en tout état de cause que devant les prud'hommes la charge de la preuve incombera aux salariés et que cela relève de l'inscription dans la loi de la logique du pot de terre contre le pot de fer, la procédure sera de facto difficilement opérante au vu des délais et des coûts qu'elle implique, cerise sur le gâteau, nous avons toutes les raisons d'estimer que cette mesure comporte en réalité plus de risque juridique pour l'employeur, qu'elle ne le sécurise à l'opposé de l'objectif des partisans de cette mesure sous prétexte de clarifier l'abandon de poste, le régime même de la démission deviennent en effet équivoques au Sénat la majorité sénatoriale a encore aggravé ce texte et le gouvernement a décidé de suivre les demandeurs d'emploi ne sont pas envisagées ici comme des citoyens ayant cotisé à l'assurance chômage, de manière à bénéficier d'une indemnisation en cas de perte d'emploi, mais comme des suspects en puissance des profiteurs qui n'aurait en rien participer à financer une assurance dont ils voudraient disposer des pour se laisser râler à la paresse, il est remarquable que les amendements durcissant les conditions faites aux personnes en recherche d'emploi ne soit basée sur aucune, je dis bien aucune étude rigoureuse donnant quelques assise ou que ce soit aux projections que traduisent les choix de la majorité et du gouvernement, c'est une certaine Vox populi qui donne le ton : ici, et certainement pas des données fiables, la voix de la majorité du Sénat, validé par le gouvernement, le choix, pardon, de la majorité du Sénat, validé par le gouvernement de sanctionner une personne ayant refusé un CDD à 3 reprises, est ainsi désastreux, j'ai cité au cours des débats, l'exemple d'une personne de 50 ans qui, à cause de la fermeture de son entreprise près perdrait son emploi après 30 ans de carrière alors qu'elle bénéficiait d'un salaire correspondant à son ancienneté, ça arrive tout le temps, tous les jours partout en France, au bout de quelques mois n'ayant pas retrouvé d'emploi équivalent à celui qu'elle a perdu arrivant en fin de droits, cette personne accepte un emploi en deçà de ses aspirations légitimes un emploi moins rémunéré moins intéressant ou peut être difficile, si bien que lorsqu'on va lui proposer un CDI, cette personne ne l'acceptera pas et la situation peut se répéter plusieurs fois avant que ne puisse être enfin saisi une opportunité permettant pour elle une forme de retour à la normale à cet âge, n'est-il pas légitime d'aspirer à disposer de temps permettant de retrouver un emploi qui correspondent à une expérience et des compétences compatible avec son état de santé. Je vous le demande, à nouveau, qui sommes-nous pour inscrire dans le marbre des dispositions qui le lui interdiront qui mettront en difficulté des gens dont nous ne connaissons pas la vie. Pour conclure, je dirais que l'on ne peut pas légiférer avec esprit de justice et souci de notre démocratie sociale en ramenant les demandeurs d'emploi à une seule et même entité, un seul et même préjugés selon lesquels il serait des personnes peu empressés à retrouver un travail et qu'il faut forcer à revenir vers l'emploi, il y aurait sans doute eu de belles choses à faire dans le cadre d'un projet de loi de réforme de l'assurance chômage pour aller vers une assurance chômage négociée par les partenaires sociaux, fondé sur un mécanisme assurantiel et dotée de financements propres ouverte à ceux qui en sont exclus aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et donc nous nous opposons à ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à madame la. Présidente : Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, une petite heure a donc suffi à mettre d'accord, le gouvernement et la majorité sénatoriale sur ce projet de loi censée permettre le plein emploi, mais dont l'objectif principal est quand même la reprise en main de l'assurance chômage par le gouvernement, l'article 1er de la loi autorise donc le gouvernement a fixé, seul et à la place des organisations syndicales et patronales, les conditions d'indemnisation de l'assurance-chômage, cette remise en cause de la gouvernance paritaire marque une nouvelle étape du processus d'étatisation de l'assurance chômage qui veut moduler l'indemnisation chômage selon la conjoncture économique, le gouvernement Modi modules ainsi la durée d'indemnisation d'indemnisation selon que la situation de l'emploi est au Vert, orange ou rouge selon les indicateurs choisis par le gouvernement, le Vert entraîne une réduction de 25 % de la durée des allocations pour l'orange, la réduction sera de 15 % et si c'est rouge, la durée de l'indemnisation est maintenu, selon les calculs des organisations syndicales cette modulation va entraîner une baisse moyenne de 25 pour 100 du nombre de mois d'indemnisation. Concrètement, un demandeur d'emploi inscrits à partir de février 2023 et qui aurait bénéficié de 24 mois d'indemnisation chômage avec les anciennes règles verra ses droits réduits à 18 mois pour les plus précaires qui pouvaient bénéficier de six mois d'indemnisation avec les anciennes règles cela passera à seulement 4 mois et enfin les seniors dont on parle beaucoup en ce moment, qui avait droit à 36 mois chuteront à 28 moi cette modulation va précariser davantage de travailleurs et aggraver les disparités géographiques, cette loi est un coup de force sur la démocratie sociale qui s'accompagne d'une remise en cause du principe d'égalité cette atteinte grave aux droits des salariés a été possible grâce à la droite sénatoriale, qui a obtenu en contrepartie de son soutien des régressions sociales majeures, les républicains ont obtenu l'encadrement de l'abandon de poste désormais les salariés qui abandonnent leur poste seront considérés comme présumés démissionnaire et par conséquent perdront le bénéfice de l'indemnisation chômage, bravo, je rappelle simplement que ni le ministère du Travail ni Pôle emploi ne dispose d'études statistiques et d'études sur les abandons de poste en France, cette disposition repose donc uniquement sur une instrumentalisation de l'abandon de poste par certains employeurs mais surtout une procédure déséquilibré pour les salariés, totalement inadapté à la réalité de la justice prud'homale, enfin, le gouvernement a accepté de supprimer l'indemnisation chômage des salariés en CDD ou en contrat de mission qui refuse de contrat à durée indéterminée, après avoir favorisé financées par des milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales le il arrive maintenant que les contrats les après avoir, je vais y arriver exonérée des cotisations sociales des contrats courts, la droite sénatoriale donc et le gouvernement pénalise pénalise aujourd'hui ça et ceux qui refusent un CDI Rob bravo le le député Marc Ferracci, rapporteur du texte à l'Assemblée, a reconnu lui-même que les abandons de poste et les refus de CDI sont décidés, c'est des situations non massive, alors pourquoi pénaliser des comportements minoritaires. Avec ce texte, vous inverser le sens même de l'assurance chômage qui considère que les salariés doivent être protégés contre la perte de leur travail, désormais ce sont les employeurs qui sont protégés contre les salariés du choix de leur contrat de travail, en conclusion, cette loi est une attaque contre les droits des travailleurs et des chômeurs qui nous donne un quand même un avant-goût des mauvais coups à venir de la part du gouvernement, qui peut donc compter sur la droite au Sénat pour conserver une majorité parlementaire les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste porte, vous le savez, un autre projet qui repose sur une véritable sécurité sociale professionnelle et pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi, je vous remercie. Si, si, madame la présidente. La parole est à monsieur Olivier nos pour le groupe Union centriste pour cinq minutes. Madame la présidente, madame, madame la ministre, chers collègues, ça lui aussi la présidente de, de, de la commission Frédéric puis ça m'a accompli ces échanges amicaux presque fraternels empreint de de vérité ça lui aussi son son énergie les discussions que nous avons eue avec Marc Ferracci, comme on dit au rugby parfois viril mais correct même un peut être un peu plus et remercié les administrateurs pour leur travail, je pense qu'on a abouti à un projet de loi équilibré le le meilleur possible, qui correspond aux réalités qu'on vit au quotidien, hein, les tensions sur le marché du travail, combien de d'entreprises ne peuvent pas répondre à tous les marchés, par manque de personnel ou de restaurants ferme plus tôt, hier encore, hein, je crois que c'est la réalité aujourd'hui et qui est la réalité française, et donc ce projet de loi est un pragmatisme, c'est pas une position morale non c'est un pragmatisme, ça correspond à à la réalité du marché du travail, il faut dans ce pays des incitations plus fortes au travail bien sûr une juste rémunération du travail, mais c'est la question de la de la valeur travail et je pense que nous avons été animée par cette question de la valeur travail tout au long de la discussion de ce projet de loi et au-delà de l'attachement à la valeur travail, quels sont nos marqueurs Mano marqueur, c'est la défense du paritarisme, c'est l'ADN du Sénat mais aussi de nos groupe UC et à LR, c'est l'idée que le paritarisme est un pilier du modèle français de de solidarité, il en va ainsi pour l'assurance chômage pour la retraite pour la protection sociale, le modèle français de protection sociale, ça n'est pas l'étatisation et puis bien sûr notre notre autre marqueur, c'est l'assurance chômage, l'assurance qui doit protéger des accidents, mais qui n'est pas là pour protéger de toutes les situations de la vie et donc à un abandon de poste, il n'a rien de choquant pour répondre que ça corresponde à une démission, c'est la réalité et que lorsqu'il y a refus de de CDI, on puisse s'interroger sur la nature de l'assurance chômage et je le dis, c'est au bénéfice des salariés parce qu'ils sont les principaux contributeurs de cette assurance, l'argent ne tombe pas du ciel, à noter aussi que la CMP a conservé l'assouplissement des règles du CDI intérimaires que la commission des affaires sociales avait introduit, nous pouvons également nous réjouir que soit maintenu l'article issu d'un amendement de notre collègue Philippe Bas qui introduit un parallélisme des procédures en cas d'indemnisation du chômage d'un ancien agent par une collectivité territoriale, nous n'avons pas oublié que le Sénat représenter les territoires et les collectivités, et puis en matière d'élections professionnelles, le sénat a introduit à l'initiative de Catherine Procaccia, un article visant à sécuriser les mesures de représentativité des organisations syndicales dans les branches de l'enseignement privé. Je m'arrêterai surtout enfin sur les dispositions relatives à la valorisation des acquis de l'expérience que j'ai tout particulièrement suivi en tant que rapporteur je salue vos propos, Madame la Ministre, sur la la VAE, le Sénat avait souhaité inscrire dans la démarche engagée par le gouvernement et par l'Assemblée nationale qui vise à donner un nouveau souffle à la VAE en la rendant plus accessible et en renforçant l'accompagnement des candidats dans cette perspective, nous avons souhaité sortir d'une approche par statut en posant le principe d'une VAE ouverte à toute personne dont l'expérience est en lien avec la certification visée, la CMP a conservé à l'Arctique quatre cet apport du Sénat qui permettra d'éviter les risques d'exclusion de certaines personnes, l'émission du GIP pour créer, pour mettre en oeuvre le service public de la VAE devront être assurés en tenant compte des besoins en qualification selon les territoires, comme nous l'avions souhaité le Sénat avait enfin introduit à l'initiative du gouvernement un article 4 bis prévoyant l'expérimentation d'une VAE dites inversée qui permettra, dans le cadre de contrats de professionnalisation de combiner formation en alternance et parcours de pour conclure sur la VAE je pense que c'est une question dont on n'a pas fini de parler, on l'a abordé, on l'aborde souvent par les aidants et les proches aidants, mais c'est bien sûr, ça les concerne, mais c'est un grand sujet, c'est la question de la formation à tous les âges de la vie, il y a la formation initiale, il y a la formation continue et là il y a la valorisation des acquis de l'expérience et je voudrais pour conclure, hein, je lisais l'autre fois qu'au Danemark, il y avait plus de 30 % plus de 50 pour 100 même parfois des gens qui se former jusqu'à l'âge de 65 ans, et au moment où on s'interroge sur les questions de de retraite et de l'emploi des seniors, hé bien je pense que la formation tout au long de la vie, c'est une grande question et que cette VAE doit permettre d'aller plus loin sur cette question de la formation tout au long de la vie, bien sûr, nous voterons ce texte parce que je crois qu'il fait oeuvre utile, je vous remercie toutes et tous. Merci, merci, cher collègue, la parole est à madame Pentel pour le groupe. Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes. Madame le président, madame la ministre, madame la le rapporteur, madame la présidente. Mes chers collègues, nous arrivons donc à la fin des discussions autour de ce projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, a pris la CMP, du 9 novembre dernier lorsque nous avons observé d'arriver de ce texte l'agenda parlementaire, force est de reconnaître que le choix des mots opérée par le gouvernement pour le qualifier était ingénieux dans l'optique de conquérir une massive adhésion ainsi qu'il peut ainsi qu'il peut donc bien s'opposer publiquement à l'aspiration au plein emploi, peu de monde, toutefois nous avons rapidement saisi qu'il s'agissait en réalité du commencement d'une série de réformes d'ampleur du marché du travail, bien que l'intention soit partagé par bon nombres d'entre nous, sur ces bancs, il aurait été préférable que nous puissions aborder ces travaux avec un peu plus de transparence sur les étapes qui vont suivre dans les prochains mois en effet, bien que nous progressions dans un contexte incertain affectant les projections économiques l'Exposition initiale d'une feuille de route claire aurait certainement suscité des débats plus serein, notamment avec les partenaires sociaux, syndicats professionnels et organisations patronales. Au-delà des considérations sur la méthode, nous souhaiterions néanmoins salué l'investissement de chacun et de chacune, ainsi que, comme l'a exprimé ma collègue Maryse Carrère en première lecture le chômage de masse ne soit plus une fatalité au sujet de la principale disposition inscrite dans l'article 1er, nous parvenons à reconnaître que cela va permettre de préserver de système d'assurance chômage pendant une période transitoire durant la caisse laquelle pardon, une phase de concertation puis de négociations sur les règles de gouvernance s'ouvrir avec les partenaires sociaux, cela octroiera une certaine agilité au gouvernement pour disposer d'une base permettant d'intégrer dans le futur décret des modulation des règles d'indemnisation, tenant compte de la conjoncture économique, mais la prudence ce que nous exprimons à l'origine sur le potentiel détricotage de la gestion paritaire du régime d'assurance chômage reste d'actualité. Toutefois, monsieur le ministre, Olivier Dussopt devant les députés, s'est engagé à ne pas modifier les conditions d'affiliation au système de l'assurance chômage et de ne pas diminuer le nombre de personnes éligibles à l'ouverture des droits et c'est naturellement une bonne nouvelle, elles aussi, la durée de 6 mois, travailler au cours des derniers 24 mois issu de la réforme 2019 est maintenu. Au sujet de la présomption de démission pour les salariés, un abandon de poste, les privant d'accéder à l'à l'indemnisation chômage, nous sommes au quotient que cette mesure répond à une préoccupation de tirer les apports du Sénat sécurise le dispositif pour que le salarié puisse contester la rupture de contrat devant le conseil des prud'hommes, il faudra tout de même être attentif à ce que le jugement prononcé sur le plus rapide possible pour que dans l'intervalle, le salarié ne soit pas totalement délaissé dans une situation précaire. D'autre part, la majorité sénatoriale aura réussi dans le cadre de groupe pour d'un compromis avec le gouvernement à mettre en place l'absence d'indemnisation pour refus de contrat de travail à durée indéterminée à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée pour nous, cette mesure est une véritable usine agace dans la mise en oeuvre risque d'être compliqué au regard d'une procédure de vérification alambiquée, le groupe RDSE se félicite en revanche de la réforme de la validation des acquis de l'expérience qui permet à toute personne d'obtenir une certification véritable diplôme grâce à son expérience, la VAE ne s'est pas suffisamment imposées dans le paysage de la formation professionnelle, or il s'agit d'un outil permettant de réaffirmer que l'acquisition de compétences techniques, dans le cadre d'une activité professionnelle et tout aussi intéressante que la validation d'une formation initiale. Pour conclure, nous partageons l'idée que les droits sociaux des travailleurs et des demandeurs d'emploi doivent au pouvoir être préservé, sous le regard attentif destin de dialogue social sanctuariser et pérenne, néanmoins, nous sommes quelques-uns au sein du groupe RDSE à éprouver un sentiment d'inachevé et à rester sur notre faim quant à la propension de ce projet de loi à répondre de manière ambitieuse aux besoins des plus exposés aux risques sociaux et en particulier le chômage, de même qu'aux besoins des secteurs d'activité qui éprouvent des difficultés de recrutement ainsi fidélité avec la tradition de liberté du vote, les membres du groupe RDSE feront des fois pluriel à cette occasion je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Chantal de scène pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

l'accord trouvé en commission mixte paritaire a permis au Sénat d'élargir l'ambition du présent texte. Nous avons tout d'abord souhaité rétablir le respect du paritarisme, mise à mal par la réforme de 2018, la loi du 5 septembre 2018 dessaisi en effet en grande partie des partenaires sociaux de leur pouvoir, selon des règles strictement défini par le gouvernement, le texte adopté en CMP prévoit donc l'ouverture d'une négociation interprofessionnelle l'année prochaine, qui portera sur la gouvernance de l'assurance chômage, ainsi que sur les conditions de l'équilibre financier du régime, le document d'orientation transmis pour la négociation invitera, par ailleurs, les partenaires sociaux. à négocier sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage issues de la réforme de 2018, il est en effet nécessaire de tirer les leçons de l'échec de cette réforme, le projet de loi a ainsi pris une direction imprévue permettant d'engager une vraie réflexion sur la gouvernance de l'assurance chômage, dans un esprit d'autres d'opposition à l'étatisation du régime d'autre part, lors de ces débats, le Sénat s'est attaché à protéger les droits des demandeurs d'emploi en garantissant que les indemnités chômage soit octroyé de manière équitable, nous avons validé et sécuriser le dispositif introduit par l'Assemblée nationale. Sur les abandons de poste qui sont présumés être des démissions en effet sauf motif légitime l'arrêt volontaire de travail ne doit pas pouvoir donner lieu à une indemnisation au titre du chômage. Nos rapporteurs ont également souhaité traiter la question des refus répétés d'offres d'emploi, la commission des affaires sociales avait prévu que ne puisse être ouvert le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage aux salariés qui aurait refusé un CDI à 3 reprises, la même année, suite à un. CDD le constat, de nombreux refus d'emploi stable à l'issue de mission d'intérim, nous avait également conduit en séance à supprimer l'indemnisation de l'intérimaire, refusant de poursuivre son activité. je tiens à féliciter nos rapporteure, Frédérique Puissat et Olivier Henno, qui ont su parvenir à un con. Promis en CMP sur ce sujet sensible, en accord avec les députés, ils ont fixé à 2 le nombre de refus ne pouvant être considéré comme acceptable, il ne s'agit pas de sanctionner ainsi l'abandon de poste ou le refus d'un CDI, il s'agit de faire respecter la nature assurantiel du régime d'assurance chômage, dans le cadre de ce régime des indemnités chômage ne peuvent s'adresser qu'aux personnes involontairement privée d'un accès à l'emploi ainsi que l'a indiqué notre rapporteure Frédérique Puissat à partir du moment où nous avons adopté ces dispositions, elle devrait, elles devront entrer en application, il vous appartiendra à Madame la Ministre, d'accompagner les chefs d'entreprises pour leur éviter une surcharge administrative de même, vous aurez la responsabilité de mettre en oeuvre le principe de modulation que nous avons souhaité inscrire en toute l'aide dont le projet de loi l'existence de nombreux emplois non pourvus et les difficultés financières du régime justifie en effet que les règles d'indemnisation soit adapté à la situation économique en cours, mais sous réserve que soit trouvé les bons paramètres de cette modulation, nous serons donc particulièrement attentifs aux conclusions que vous rendrez sur ce point, le 21 novembre prochain comme l'indique son intitulé le projet de loi vise à atteindre le plein en plein emploi, je tiens à souligner les apports du Sénat en ce sens qu'il s'agisse par exemple des précisions sur l'expérimentation du CDD multi- remplacements ou encore du déplafonnement de la durée du CDI intérimaires concernant la problématique des contrats courts, nous regrettons que la réunion en commission mixte paritaire n'est pas permis de recentrer comme nous le souhaitions le disponible, le dispositif de bonus-malus sur les cas de contrats précaires initialement invité à un moment où les charges pèsent particulièrement sur les entreprises, il nous semble également nécessaire de revoir le taux de leur taxation, ce que n'ont pas souhaité les députés de la majorité, enfin, afin de renforcer l'accès à l'emploi, le gouvernement a souhaité créer un service public de la validation des acquis de l'expérience lors de l'examen du texte, nous avons décidé de l'ouvrir à tous supprimons les aléas de statut et simplifiant davantage les procédures, en conclusion, le projet, le projet de loi n'est pas un texte décisif pour atteindre le plein emploi, son ambition première était d'ailleurs d'assurer la continuité du régime d'assurance chômage au-delà de ce mois de novembre mais le travail de nos rapporteurs que je tiens à nouveau à féliciter a permis des de sauver ce texte en prônant le respect du travail, la protection de notre régime d'assurance chômage et la défense du paritarisme aussi le groupe Les Républicains votera-t-il ce projet de loi, je vous remercie. Merci alors. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi ordinaire dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire et modifié par les amendements de la commission, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains et le groupe Union centriste sur l'ensemble du texte, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Alors résultat du du scrutin Nombre de votants : 343 exprimés 333 pour 242 contre 91, le Sénat a adopté. La parole est à madame Guilaine Pentel pour une mise au point au sujet d'un vote. lors du scrutin numéro 55 portant sur l'ensemble de la proposition de résolution portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France et l'amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre, le groupe du RDSE, n'a pas pris part au vote alors qu'il souhaitait voteraient pour.